La séance est reprise, mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunis en fin d'après-midi sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observation. Je considère ces conclusions comme adopté. Nous reprenons la discussion. Du projet de loi rejeté par l'Assemblée après engagement de la procédure accélérée de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Mes chers collègues, et il nous reste 68 amendements à examiner sur ce texte, mes chers collègues, et Monsieur le Ministre. Il ne vous a pas échappé que notre ordre du jour, a prévu que nous devons achever l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques ce soir. Même tard. En effet, l'examen du projet de loi relatif à l'accès à l'accélération de la production d'énergie renouvelables débutera demain matin à 10 heures 30 avec au menu 669 amendements, nous ne devrions pas en principe prolonger notre séance de ce soir, au delà de une heure 30 pour ne pas décaler l'ensemble de l'ordre du jour avec les, les, les temps de d'observation j'observe donc chacun à respecter dans la mesure du possible, une certaine concision dans ses interventions. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 62 au sein de l'article 3. Et c'est un amendement du gouvernement Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais m'attacher, être très concis, c'est un amendement de rétablissement de la trajectoire qui avait été proposé dans le cadre du projet de loi texte initial du gouvernement et donc on se souvient que les amendements qui ont été adoptés en commission ont prévu une accélération très rapide du rythme de maîtrise de la dépense publique avec un Quantum d'économie qui nous semble objectivement trop élevés à court terme et donc c'est un un moment qui propose de rétablir la trajectoire initialement proposé par le gouvernement. Monsieur le rapporteur général l'avis de la commission. L'avis est défavorable, je sais pas si l'amendement, enfin, je suis un peu surpris. Par les certains mots employé par le ministre-parce que dire qu'un amendement sénatorial état d'amendement trop rapide pour le rétablissement de la trajectoire je crois pas que ce soit le cas, cette l'amendement du bon rythme qui permet à la France de retrouver la bonne trajectoire et Monsieur le Ministre d'ailleurs de le faire comme un certain nombre de nos partenaires européens. Il ne va pas d'observation, je mets le convoi cet amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 77 présenté par le rapporteur général. Correction d'une erreur matérielle pardon. Gouvernement. Très rapidement, c'est un amendement de mise en cohérence, sur le niveau de la dette liée à la trajectoire qui a été adopté, j'ai dit que nous ne partagions pas intégralement cette trajectoire mais par cohérence, parce que j'aime les tableaux bien rempli les textes bien écrits, je donne un avis de sagesse.

Monsieur le pense qu'il y a une omission, alors c'est encore un tableau, mais on va y arriver mais nous considérons que c'est un peu une quand même une bombe à retardement, puisque les émissions de la dette indexée sur l'inflation, c'est quand même une question importante, fin 2021, l'encours des titres indexés émis par l'État s'élever à 236 4 milliards dont 167 7 6 milliards indexée sur l'inflation de la zone Euro, pour un total d'encours de la dette négociable de l'État de 2145 milliards et les géants sur lesquels on est les volumes 72 % des obligations indexées leçons sur l'indice des prix à la consommation de la zone Euro, alors même que l'inflation est un plus forte au sein de la zone Euro 10 % qu'en France, à peu près 6 2 pour la seule année 2021 les titres indexés ont renchérit la charge de la dette de huit virgule 8 milliards, donc c'est pour vous dire le souci qu'on a aussi sur la dette, donc nous estimons que le phénomène mérite d'apparaître clairement dans la programmation de sorte à maintenir une prési visible une prési visibilité sur la charge de la dette à moyen terme et j'ai ressorti à INA quatre le tableau après la 16ème ligne où là nous proposons d'insérer la part d'obligations assimilables au Trésor indexés sur l'indice des prix de la zone Euro. C'est une demande de de retrait en fait le tableau, c'est plutôt une présentation des objectifs et non pas une présentation extrêmement précise et minutieuse d'un tableau qu'il faudrait mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, donc un avis de retrait. Ministre. Très rapidement, c'est un amendement qui propose de décomposer la dette entre les OAT, les OAT indexées sur l'inflation, c'est un moment qui est pour moi satisfait puisque toutes ces informations sont disponibles dans le rapport sur la dette, dont les données ont même été renforcées par le législateur dans la nouvelle loi organique des lois de finances, donc c'est satisfait puisque toutes les informations, vous demandez sont disponibles dans le rapport annuel sur la dette il y même maintenant dans le cadre du PLF, un débat sur la dette peut être un point simplement rapidement sur la question des OAT indexées sur l'inflation, parce que c'est un débat qui revient souvent, moi ce que je veux dire et ce que je veux rappeler, c'est que tous les pays du G7 et maintenant la quasi-totalité, je crois, des pays de l'OCDE ont des obligations indexées sur l'inflation depuis d'ailleurs plusieurs décennies que c'est une part de nos obligations qui est somme toute assez réduite qui est autour de 10 % que nous le faisons parce que c'est un type de titres qui est recherché par une partie des investisseurs qui veulent se couvrir du risque inflationniste, il y a quand même une contrepartie à ça, c'est que les OAT émises le sont à un taux très nettement inférieur au taux pour des OAT classique, en l'occurrence sur les OAT indexées à 10 ans nous empruntons avec un taux de 0 15 contre 2 7 % pour un emprunt classique et par ailleurs, le coût de ces OAT indexées sur l'inflation doit s'apprécier sur l'ensemble du cycle économique de l'emprunt, et pas uniquement sur quelques années où il y aura une inflation importante, mais voilà, je voulais rappeler ces faits là parce que c'est un sujet et légitimement qui revient beaucoup dans le débat dans une période de forte inflation. Donc : demande de retrait ainsi. Ce Savoldelli oui merci Monsieur le Président, moi je doute pas de votre sincérité, donc si vous dites que c'est dans le document, c'est dans le document. Donc je le retiens entendu merci collègue et donc ils nous votons sur l'article 3 maintenant. évidemment. La commission s'est prononcée, le gouvernement aussi, qui est pour l'article 3. Contre. Il est adopté, nous arrivons à l'article IV avec un amendement de suppression de monsieur Savoldelli numéro 29 monsieur le président, Monsieur le Ministre, nous proposons en effet de supprimer cet article parce que nous considérons que la politique ne doit pas peser uniquement sur un effort en terme de dépenses, mais que nous pourrions aussi envisager d'utiliser un levier fiscal vous dites depuis tout à l'heure, Monsieur le Ministre, que votre choix n'aide pas augmenter les impôts, mais je crois que le débat ne réside pas sur le fait de savoir s'il faut augmenter ou pas les impôts, comme si les impôts étaient quelque chose d'indéfini qui pesaient de la même manière, sur tout le monde, mais qu'il y a besoin de d'abord prendre en compte les richesses créées dans le pays et de faire un un effort de redistribution, la la trajectoire qui est proposé correspond en fait à un recul de la puissance publique puisque ça nous ramènera à un niveau de dépenses par rapport au PIB qui serait équivalent à celui de 1984 alors que, pour ne citer que cette évolution, la population a crû de 11 millions de citoyens, on ne peut donc évidemment pas raisonner de la même manière, et donc il nous semble utile de porter dans ce débat que les efforts ne doivent pas uniquement porter sur la réduction des dépenses, mais sur comment on va chercher des recettes nouvelles, et je crois que c'est un débat que nous devrions les uns et les autres engagé. Si monsieur le rapporteur général. C'est un avis sans surprise défavorable puisque j'ai bien exprimé que nous pensons, au moins une partie de cette assemblée, qui me semble majoritaire qu'il nous faut faire des efforts, y compris sur le sujet de la dépense publique, raison pour laquelle l'avis est défavorable. Monsieur le Ministre. Même avis pour les mêmes raisons. Je mets aux voix l'amendement vingt-neuf avec des le double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est pas adopté amendement numéro 63 du gouvernement Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, c'est toujours dans la série d'amendements de rétablissement, en tout cas où je tente de rétablir des dispositions du texte initial du gouvernement, en l'occurrence ici, s'agissant de l'effort structurel et donc voilà dans la même logique que les autres amendements de rétablissement que j'ai proposé depuis tout à l'heure, c'est un amendement qui vise à revenir vers la proposition initiale, porté par le gouvernement dans ce projet de loi. Monsieur le rapporteur général. Et pour ma part, je propose de maintenir l'effort proposé par la majorité sénatoriale. D'accord, un avis pardon défavorable. On pouvait le deviner donc sur l'amendement 63 du gouvernement faisant l'objet d'un avis défavorable de la commission, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, il n'est pas adopté donc vote sur l'article IV qui est pour. Contre. Il est adopté, je mets aux voix, l'article 5 sur lequel il n'y a pas d'amendement même vote.

Merci monsieur le Président, au total, ce seront 392 milliards d'euros de recettes fiscales qui ont été supprimés de cadeaux fiscaux octroyés en 10 années pour le quinquennat qui s'ouvrent, ce seront 7 milliards par an à compter de 2023 soit 35 milliards sur le quinquennat 5 milliards par an à compter de 2024 soit 35 milliards sur le quinquennat 5 milliards par an à compter de 2024 soit 20 milliards sur le quinquennat un milliard 5 par an à compter de 2025 soit 20 milliards sur le quinquennat un milliard 5 par an à compter de 2025 soit 4,5 milliards sur le quinquennat dans un contexte de crise économique, écologique et sociale, le choix, ce choix est celui de l'irresponsabilité budgétaire et de l'abandon des territoires et des populations qui en ont le plus besoin, c'est pourquoi l'Euro, socialistes, écologistes et s'y oppose fermement. Entendu amendement numéro 15 présenté par Messieurs de pertes de ressources alors que nous sommes confrontés à une triple crise sociale climatiques et économiques, c'est une mesure de désarmement de l'État qui va à contresens des défis qui s'annoncent en tous les cas de notre capacité à les assumer cet article ne constitue en aucun cas pour nous un outil qui prépare l'avenir, ils nous condamnent plutôt à une inaction au détriment des collectivités locales et des foyers dans le besoin, nous demandons donc la suppression de cet article 6. Et Monsieur Savoldelli. C'est pas mal, c'est fait, mais on apprend aussi que la dans l'actualité, le gouvernement, ils l'entendent réduire de 16,5 milliards la fiscalité sur le quinquennat en du en déduisant des mesures nouvelles et la facture serait d'au moins 7 milliards pour 2023, moi j'ai regardé ces suppressions de la contribution à l'audiovisuel public, coût 3 2 milliards. On les aura pas pour les recettes de l'État, la baisse de la première partie de la CVAE coûtera 4 1 milliard et on soustrait encore pour l'État, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ça coûtera juste 6 2 milliards et enfin la suppression définitive de la taxe d'habitation pour les plus riches qui coûtera de 8 milliards supplémentaires voilà je je ne vais pas vous et plus long sur la liste, mais c'est une mauvaise liste pour l'État. que c'est des recettes en moins quoi. Voilà, je ne vais pas développer plus loin le propos, mais nous on a essayé, j'ai essayé, ce matin encore, aux commissions des Finances de poser la question de recettes plus importante pour l'État, pour développer des politiques publiques, ce qui n'est pas le cas dans cet article, bien évidemment. Monsieur le rapporteur général, la vie, sur les trois amendements. Ce sera évidemment personne n'est surpris un avis défavorable je pense que le fait de d'avoir une disposition de ce type d'abord c'est obligatoire dans le cadre d'une loi de programmation, en vertu de la LOLF et puis je pense que les prélèvements obligatoires doivent diminuer finalement en proportion du PIB, en tous les cas en France et mais par contre pour tenir compte de l'évolution de l'impératif d'équilibre des comptes publics, il me semble qu'il faut fixer un plancher programmatique à cette baisse de manière à pouvoir tenir la trajectoire que nous, nous ce Oui c'est un avis défavorable, aussi, au fond, c'est des amendements de suppression, c'est vrai que les choses sont assez claires, c'est vrai que si vous êtes pour augmenter les impôts, il faut voter ces amendements de suppression, pour le coup, les choses sont très claires : nous on veut effectivement continuer à les baisser, c'est ce que prévoit cet article 6, j'entends que vous ayez une opposition et vous l'avez eu l'occasion de le dire dans un précédent débat, à la suppression de la contribution à l'audiovisuel public qui a été adopté pour les raisons que vous aviez évoqué sur la question de la CVAE je l'entends aussi pour les raisons que vous l'aviez évoqué pour le coup, plus de perplexité, c'est sur la 3ème mesure que vous avez cité pour la critiquer, c'est l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Pour le coup, on est vraiment sur une mesure de soutien aux classes moyennes et même aux catégories vont dire modeste qui payent l'impôt sur le revenu, si on ne prenait pas cette mesure, qui effectivement coûte de 6,4 milliards d'euros, ça équivaudrait à une augmentation de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et pour les Français qui bossent, qui galère et qui verraient leurs impôts sur leur leur impôt donc là pour le coup sur sur ce point là, je ne, je ne comprends pas votre position en tout cas c'est un avis défavorable et pardon je, je, je peux quand même indiqué parce que vous aviez dit pourquoi est-ce qu'on s'interdirait d'augmenter les impôts, et évidemment faut jamais s'interdire de rien, en tout cas, nous on a donné une garantie, c'est que tant que nous serons responsabilités, c'est-à-dire un engagement du président de la République, non seulement on n'augmentera pas les impôts, mais on continuera à les baisser, on a beaucoup fait de comparaison européenne depuis le début de cette journée pour expliquer que la France revenait plus tard que les autres sous les 3 % s'il y a un point sur lequel on est quasiment champion d'Europe, c'est quand même toujours sur les prélèvements obligatoires. On est le 2ème pays européen après le Danemark en terme de prélèvements obligatoires, ce qui justifie quand même de notre point de vue de continuer les baisser. Je peux donc mettre aux voix à ces trois amendements identiques de suppression. Qui est pour. Qui est contre.

Merci monsieur le président, il s'agit là d'un amendement de de repli, hein, qui vise à acter le le principe d'une stabilité des recettes fiscales pour le quinquennat qui s'ouvre après 5 années de baisse, centrée sur les plus aisés et les grandes entreprises, je veux pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au moins pour la la suite mais il me semble que la la réponse du ministre à l'instant été éclairante, néanmoins il n'est pas, il n'est pas raisonnable, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, même la la Cour des comptes a a pointé ce ce risque, hein, il n'est pas raisonnable de poursuite de la sorte un désarmement fiscal qui se traduit à la fois par le creusement du déficit et de la dette et par les coûts budgétaires brutales pour les politiques publiques et en particulier à destination des des plus fragiles, donc pour le moins, au moins, ne ne pas rebaisser les impôts pour les années qui viennent. Monsieur le rapporteur général. Alors, sans surprise, un avis défavorable, on a eu l'occasion à plusieurs reprises et depuis un certain temps d'ailleurs dans cet hémicycle de rappeler le niveau élevé des prélèvements obligatoires de toute nature en France on sait. Que ça pèse sur la compétitivité de nos entreprises, ça pèse aussi parfois sur le budget des ménages et pas que les plus aisés sur en tous les cas une partie de l'argumentation à l'instant sur l'indexation de l'impôt sur le revenu, il faut faire attention parfois le, le mieux est l'ennemi du bien et donc un avis défavorable sur votre amendement. Monsieur le Ministre. Même avis pour les mêmes raisons. Je me vois cet amendement numéro IV qui est pour. Quelles sont les collègues qui sont contre. Abstention : il est adopté, il est, pardon, il a écarté excusez-moi et non je fais voter sur l'article 6 qui est pour. Contre. Article 6 est adopté l'article 7 nous avons un premier amendement numéro

même si a la remise d'un rapport tout ça n'exonère pas le pouvoir de s'affranchir de ces délais, c'est un débat qui a été par exemple un article qui avait été rejeté à l'Assemblée nationale, juste un point de repère le chiffrage des dépenses fiscales à une fiabilité limitée, on peut peut-être le reconnaître ensemble, j'ai regardé sur les 465 dépenses fiscales recensées en projet de loi de finances pour 2023 56 n'ont pas de chiffrage, au titre de 2021. Dernière exercice clos parce que leur coût n'a pas pu être déterminée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vigilant quand même et je pense que le délai de 2 ans me paraît correct pour avoir un examen commun aussi bien exécutif que les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat sur toute fixation de de de niches fiscales, qu'on soit d'accord ou pas avec la niche fiscale, je pense que 2 ans, ça permet d'être évalué et d'être apprécié merci. Ce rapporteur général. Il est en discussion commune le temps pour moi avec un amendement 52 présenté par Madame Paoli-Gagin qui est défendu par Monsieur. bah, l'amendement va exactement dans le sens inverse, il propose-lui de rallonger à 5 ans la durée de prolongation pour les raisons hein, je rejoins ce qui a été dit, c'est compliqué de calculer le coût mais c'est encore plus calculs compliqués qui appuie le coup sur deux ans donc l'amendement propose lui d'étendre à 5 ans pour avoir le temps d'examiner la pertinence des des dépenses mise en en place.

d'autres collègues, propose 5 et nous avons en commission choisi trois 3 ans donc je je propose de rester à l'heure à la fois un petit trait d'humour, mais peut être sérieusement je pense que 2 ans pour procéder à l'examen des dépenses fiscales et je partage l'avis de notre collègue Savoldelli, c'est-à-dire le fait de dire on doit regarder de plus près les dépenses fiscales, une à une, mais le faire trois ans nous est apparu comme un délai raisonnable, parce que d'abord, je le dis, un certain nombre de dépenses fiscales ne sont même pas évaluer et le fait de le faire chaque année avant les évaluer avant les 3 années ça permet justement d'avoir une meilleure connaissance et de s'astreindre à ce travail indispensable pour ensuite en tous les cas, c'est Simon veut regarder si ces dépenses fiscales sont utiles et doit être conservé trois ans paraît un délai raisonnable 2 ans est vraiment trop court et 5 ans alors pour le coup, beaucoup trop long. Donc à double avis défavorable. Oui, d'abord, c'est important de souligner la qualité de ce dispositif qui permet d'avoir une évaluation à bornage dans le temps des niches fiscales, c'est une introduction, il me semble, la loi de programmation des finances publiques 2018, 2022 qui est prévu, effectivement, tous les 4 ans dans le texte initial, on a repris 4 ans aussi, j'ai vu que la commission des finances avait adopté un amendement pour amener à 3 ans, ce qui me semble effectivement c'est plus exigeant, d'un point de vue du contrôle du Parlement, mais c'est aussi l'objet de ce texte et donc moi je suis plutôt favorable, ouvert à ce choix qui a été fait par la commission des finances, donc voilà, je demanderai je donnerai un avis défavorable, 2 ans, c'est vrai que c'est, c'est trop peu, d'autant que l'impact d'une niche fiscale, enfin, par définition, elle produit son impact sur le bénéficiaire déjà sur l'année suivante au moment des impôts et donc vraiment 2 ans c'est trop court 5 ans c'est-à-dire rallonger le délai qui existe aujourd'hui, je, je pense que ça prive un peu le le Parlement d'un contrôle plus fréquents des dispositifs donc avis défavorable sur ces amendements. Alors nous commençons par l'amendement quarante-quatre, présenté par Monsieur Savoldelli avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Donc il n'est pas adopté quant à l'amendement 52 de Madame Paoli-Gagin avec double avis défavorable aussi qui est favorable, qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté, non plus, donc nous pouvons voter sur l'article 7. Qui est pour, contre. Il était adopté, après l'article 7 nous avons un amendement pourtant addict articles additionnels qui est présenté par Monsieur de La Haye et il y a un amendement identique du gouvernement simplement neutre. Bernard. Collecte de lait et seul signataire et il n'est pas avec nous, à l'instant, donc on va examiner seulement l'amendement 64 du gouvernement. Merci monsieur le Président, c'est dommage, j'aurais bien aimé dans cette soirée, avoir un amendement identique au gouvernement défendu, pas de chance, l'auteur n'est pas là mais j'imagine son groupe sera solidaire de son amendement et votera l'amendement du gouvernement, c'est un amendement qui propose de rétablir une disposition qui est issu. Du texte. Comment de l'Assemblée, mais qui est le texte du gouvernement : c'est une disposition qui avait été proposée, pardon, par un parlementaire à l'Assemblée nationale, comme le texte a été rejetée, une fine et par le Parlement, c'est le texte initial du gouvernement qui arrivent ici, mais qui propose d'introduire un ratio entre eux une baisse du ratio entre dépenses fiscales et budget général à horizon de 5 pour 100, horizon 2028 l'objectif, c'est de dire qu'il faut baisser les niches fiscales, réduire les niches fiscales baisser la dépense fiscale dans notre pays et donc on se donne un objectif à horizon 2020, 28 de baisser de 5 % le ratio entre la dépense fiscale et le budget général, c'est un député Mathieu Lefèvre je crois qu'il avait proposé cet amendement qui avait été adopté par la commission des finances, puis ensuite, je pense en séance qui avait été confirmés. Comme le texte a été rejetée, il n'arrive pas ici dans le texte initial comme ça nous semble être une bonne idée parce que c'est de bonne gestion que de réduire la dépense fiscale dans notre pays, on propose de réintroduire, comme le sénateur de l'lait. L'avis de la commission de suivi rapporteur général. L'avis est défavorable, je vais donner quelques dans l'explication, effectivement de l'amendement était présenté par Mathieu Lefèvre et me semble-t-il, le rapporteur général de la commission des finances, alors on a un petit problème de méthode qui n'est pas tout à fait anodin puisque l'objet mentionné, effectivement, le pourcentage de. Dépenses fiscales par mission budgétaire mais la rédaction vise l'ensemble des crédits budgétaires toutes missions confondues, or, à ce stade, ces crédits ne sont pas précisément définis et ce qu'il s'agit en fait de la totalité des crédits du budget général ou des crédits sur le nouveau périmètre de l'État ou d'une autre définition, en second lieu, l'amendement n'aurait de toute manière qu'une portée mineure puisque si on considère la totalité des crédits du budget général, c'est-à-dire un peu plus de 560 milliards d'euros, le rapport prévu par cet amendement serait laissons le mes calculs, de 15,9 % actuellement et donc la diminution de 5 pour 100 que prévoit cet amendement signifie que le rapport passerait non pas à 15 9 % mais à 15 1 % dans cinq autant le dire, une évolution à peine perceptible et puis si on regarde entre 2002 2023, le montant des dépenses fiscales devraient diminuer de 5 milliards d'euros, soit plus de 5 % sur un seul exercice alors pourquoi, a rapporté le montant des dépenses fiscales au crédit et non pas aux recettes, je m'en étonne c'est une mesure qui me paraît finalement entre illusoire et superfétatoire, d'où la demande de retrait. Monsieur le Ministre. Non, peut-être juste pour répondre au rapporteur général, c'est bien sûr l'ensemble des missions du budget de l'État. Je suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que ça aurait un impact mineur puisque par définition le budget général de l'État va continuer à augmenter. D'ici à 2000 28 et donc la baisse du ratio se fait par rapport aux niveaux aujourd'hui sur un budget qui va continuer à augmenter, donc ça aurait un impact, mais si je suis votre logique de ce que vous m'avez répondu sur l'article 23 ans, j'ai dit qu'il n'aurait probablement pas être activée parce qu'on faisait confiance aux collectivités locales : vous m'avez dit ben alors si c'est pas si ça a pas d'impact majeur, pourquoi le faire, j'ai envie de vous retourner l'argument si vous considérez que c'est superfétatoire, pourquoi ne pas le voter ça envoie un signal qu'il faut réduire la dépense fiscale dans notre pays et je crois qu'on est très nombreux à partager cet objectif. Je n'ai pas de demande d'explications de vote, donc je vais soumettre. L'amendement 64 du gouvernement. Avec avis défavorable de la commission qui est favorable, qui est pour.

Qui est contre. Il n'est pas l'adopter. Sur l'article 8, j'ai une demande de parole de monsieur Marc Laménie, qui a la parole. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, le président de la commission des finances sur le rapporteur général, quelques mots concernant cet article 8 qui fait partie du rapport, je parle sous l'autorité des collègues, c'est un document qui fait plus de 300 pages et concernant cet article 8 il consiste au plafonnement des taxes affectées les recettes fiscales en particulier cette fiscalité affectée représente un montant important qui s'élèverait en 2023 à 3 sont à plus de 366 milliards d'euros pour mémoire en 2017 ce montant s'élevait à 259 milliards d'euros, soit une augmentation significative de plus 40 % cette répartition des 366 milliards d'euros il y a 242 milliards environ d'euros affectés à des organismes de Sécurité sociale, la CSG et la TVA a fait n'affecté pour le secteur local se s'élèverait à 58 milliards d'euros, collectivités territoriales, groupement établissements locaux et organismes consulaires, les organismes d'État administration centrale : opérateurs, établissements publics nationaux à hauteur de 43 milliards d'euros et les autres bénéficiaires dont les associations pour un montant de vingt-trois milliards d'euros à noter un lien qui doit exister entre la taxe et l'organisme bénéficiaire le montant versé au titre d'une affectation de taxe doit être plafonnée pour chaque organisme bénéficiaire limitation du plafond en fonction du rendement prévu le dispositif proposé au niveau de la commission des finances, c'est le plafonnement qui présente un Avantage pour contribuer. Ah, la transparence, notion de transparence sur le recours aux taxes affectées, soulignant que mon vote favorable à cet article, je vous remercie. Très bien. Et donc je mets aux voix, l'article 8 il y a-t-il des voix pour. Contre. L'abstention, il était adopté. Après l'article 8 un amendement un article additionnel proposée par le gouvernement, l'amendement 65, monsieur le ministre. Oui, c'est un amendement de rétablissement d'une disposition adoptée à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Pierre Cazeneuve qui propose la création d'un d'une programmation pluriannuelle des moyens de la transition écologique ça nous semblait être une mesure utile qui est d'initiative parlementaire et pour ces raisons, on propose son rétablissement. Monsieur Bruillet vous avez un amendement en discussion commune. C'est un amendement identique j'ai j'ai entendu le désarroi du ministre devant le rejet de tous ces amendements bah j'espère comme lui à avoir ce soir un amendement entendu avec cette volonté de créer une loi de programmation par non pluri-des financements la transition écologique, nous avons des objectifs nationaux et sectoriels clair en matière de transition écologique, mais sans les financements publics afférents, qui sont pourtant le pilier de la concrétisation de ces objectifs, ils ne sont pas inscrits dans un cadre législatif permettant de les programmer dans le temps long, c'est la raison pour laquelle nous proposons cette création qui donnera aux entreprises, aux ménages, aux investisseurs et aux collectivités territoriales une meilleure visibilité sur les volontés politiques de notre pays dans le domaine de la transition énergétique, j'avais entendu en commission que cet amendement pouvait prospérer, je souhaite que ce soit le cas, ce sera une façon de montrer la volonté du Sénat de renforcer cette exigence de transition écologique. Entendu, monsieur le rapporteur général. Notre collègue Daniel Breuiller, il a pas tout à fait bien entendu. Mais je vais ajouter par anticipation à la discussion commune des amendements 65 et 16 l'amendement 17 qu'il va présenter ensuite puisque c'est le dix-sept, sur laquelle je rends un avis de sagesse et sur les 16 65, une demande de retrait, je m'explique : l'amendement 17 qui arrive, prévoit que, effectivement, c'est la programmation inclut les moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs, tandis que les amendements 16 et 65 prévoit une loi séparée compatible avec la loi énergie-climat qui fixe des priorités d'action, je dis bien d'action de la politique de transition écologique et des moyens, sans préciser lesquelles, qui lui sont consacrés, je ne suis évidemment pas hostile sur le fond, hé bien au contraire à ce que les moyens de la politique de transition écologique soit prévu par une loi de programmation, je ne suis pas sûr néanmoins que les lois de programmation des finances publiques, soit le le lieu où le vecteur le le le plus approprié pour prévoir des dispositions de nature sectorielles, raison pour laquelle j'ai choisi la vie de rendent de la vie de sagesse sur l'amendement 17. Monsieur le ministre, vous avez mis le je suppose un avis favorable à l'amendement qui est identique au vôtre. Oui, j'étais même en train de me dire que, pour nous donner le plus de chances possible, j'étais prêt à retirer l'amendement du gouvernement au profit de l'amendement du sénateur brouillé, ce qui nous donnera plus de chances que l'amendement puisse être adopté, j'imagine, pour une partie de l'hémicycle de voter l'amendement de Monsieur Bruillet, plutôt que de celui du gouvernement, donc je retire mon amendement au profit de l'amendement numéro 16. Après cet effet de séance réussi je je peux mettre aux voix l'amendement cessent de Monsieur avec un avis défavorable de la commission, mais un A Vif implicitement favorable du gouvernement qui est pour.

après l'article 8 toujours, il a cet amendement dix-sept auquel il vient d'être fait allusion et donc je laisse monsieur Breuiller le préciser. Le le rapporteur général a presque défendu mon mon amendement et je remercie le le le ministre et c'est un grand moment dans cet hémicycle que de voir à quel point nos idées progressent, l'amendement dix-sept vise à ce que la politique énergétique nationale intègre réellement des moyens financiers pour permettre de réaliser les mesures ambitieuses en matière de lutte contre le dérèglement climatique, avec notamment la PPE et la baisser la France s'inscrit dans une trajectoire de neutralité carbone et une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050, il serait davantage pertinent de se fonder sur des moyens chiffrés, concrets, sans cela, il nous sera impossible d'étudier l'avancement des trajectoires, ni de nous assurer de l'atteinte de ces objectifs, définir des objectifs non rend tout simplement la loi, la plupart du temps in opérationnel, voilà l'objet de cet amendement 17. Vous avez tout dit, monsieur le rapporteur général, monsieur le Ministre. je vais donner un avis favorable à l'amendement du sénateur brouillé parce qu'on n'a pas réussi sur l'amendement précédent, ça serait dommage de ne pas sortir avec un geste non mais en faveur de la planification écologique et de la programmation de nos investissements en la matière, je pense qu'on est très nombreux à partager cet objectif et donc je je donne un avis favorable. Il y a pas de demande d'explications de vote, donc je mets aux voix l'amendement 77 pardon de monsieur voyez avec avis de sagesse de la commission et l'avis favorable du gouvernement qui est pour.

Qui est contre. Oui l'et a plus de vraiment de doute, donc il est adopté. Donc, cet article additionnel est adopté et nous passons à l'article 9 sur lequel nous avons à l'amendement 53 qui est présenté par Monsieur qui a pu. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement de notre collègue Paoli-Gagin qui propose, contrairement à ce qui est indiqué, cette année, ça n'est pas un amendement de repli qui propose de limiter la hausse des dépenses de l'État à 1 % par an par rapport au niveau des dépenses de 2023. Monsieur le rapporteur général, qui représentait une trajectoire entre moins un et moins 2 % par an en volume, compte tenu des prévisions d'inflation quand j'entends le ministre dire que déjà c'est presque la purge. Je pense qu'il faut faire attention, monsieur le sénateur, en tous les cas, je vous invite non pas instamment mais gentiment plutôt une position de retraite. Le ministre. Oui, je veux remercier à la sénatrice Paoli-Gagin et le sénateur qui a pu, de remettre dans le débat, cette question de la maîtrise de nos dépenses publiques, en l'occurrence c'est vrai que là ça fait un rythme encore encore plus fort que ce qui est proposé, ce qui, voilà ce qui objectivement ne nous semble pas atteignable, moi je veux quand même rappeler les chiffres que j'ai donné, c'était avant la pause du dîner, augmentation de la dépense publique. Toutes administrations publiques confondues.

ce qu'on propose dans la loi de programmation des finances publiques, le texte initial du gouvernement pour les 5 ans qui viennent, c'est 0 6 % donc c'est dire l'effort le plus important de maîtrise de la dépense publique depuis au moins 15 ans dans la copie, qui a été adopté par le Sénat, c'est 0 1 % objectivement, il faut toujours, on en parlait avec le rapporteur général, il y a quelques jours, viser la lune visé en tout cas le plus haut possible pour atteindre le plus haut possible, ça nous semble pas objectivement atteignable, sauf à couper vraiment massivement et drastiquement dans nos services publics, ce qui ne sont pas souhaitables, en tout cas c'est important d'avoir ce débat donc merci de l'avoir proposé. Donc je le mets au revoir monsieur. Du coup, compte tenu de ce double avis et cette demande insistante de retrait de la commission, je je le retire. Entendu donc nous passons à l'amendement 66 du gouvernement. Oui, c'est un amendement qui supprime hein. Ajout qui consiste à demander la décomposition de la norme, mais en fait cette demande de décomposition est déjà satisfaite et donc pour ces raisons, c'est une proposition de suppression. Ce que le texte initial du présent article prévoit déjà que la présentation du périmètre des dépenses de l'État sera précise et détaillée dans l'exposé général des motifs du projet de loi de finances et tous les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances présente déjà la décomposition du périmètre des dépenses de l'État, dont ça nous semblait vraiment superfétatoire que d'ajouter cette décomposition. Monsieur le rapporteur général. des motifs du PLF mais la présentation de ce périmètre faites dans l'exposé général du PLF pour 2023 se limite en fait à la définition du périmètre sans aucune donnée chiffrée, autre que le total de 480 milliards d'euros, il est donc à mon avis, étrange que le gouvernement s'oppose à une demande aussi simple, qui répond à un objectif simple de transparence des données budgétaires, d'où l'avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement du gouvernement numéro 66 avec avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté nous en venons au vote sur l'article 9. Qui est pour.

Merci monsieur le président, dans l'article 10 la stabilité globale des emplois nets de l'État entre 2023 2027 alors que les besoins d'intervention de la puissance publique sont croissant cette démarche à Paris inappropriée. Et elle conduirait inéluctablement, le gouvernement a déshabillé telle administration pour habiller, tu es à l'autre en fonction de la de la gravité des situations sociales, le groupe le groupe CR est fermement opposée à cet objectif de stabilisation des emplois et propose donc la suppression de cet article par le biais de cet amendement. Pour le groupe communiste, c'est madame brûlant qui présente l'amendement 31. Oui, en complément des arguments qui viennent d'être développé d'abord avec un grand esprit positif, je voudrais saluer. Un article qui est bien moins pire que celui de la précédente loi de programmation puisqu'il était question de supprimer 50000 emplois dans la précédente, il y avait même des esprits fous qui à l'époque, pensé qu'on pouvait supprimer jusqu'à 120000 emplois dans la fonction publique, la crise et les crises sont passés par là, et un certain nombres sont revenus à la raison, mais comme cela vient d'être dit, non seulement on ne peut pas prévoir à l'issue des crises que nous venons de vivre, quels seront les besoins dans tous les domaines de l'État, et dans ces opérateurs, mais en plus il y a un certain nombre de lois de programmation Mike qu'on a examiné, il y a. Quelques temps la loi de programmation sur la recherche, la loi de programmation militaire qui crée des emplois, alors un autre sens souvent insuffisamment, mais qui ont créé quelques-uns et donc pour rester dans cette trajectoire de stabilité si on ancrée dans certains secteurs, par définition, il va falloir en supprimer dans d'autres et c'est quand même d'abord dangereux et même très très compliqué de le faire comme ça à l'aveugle, au moment où nous sommes, je rappelle que nous avons voté à l'unanimité, ici une une proposition de loi encadrant les recours au cabinet conseil qui proposait notamment de re-internaliser un certain nombre de compétences dans l'État, ce qui semble là aussi contradictoires avec un tel objectif, c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. L'avis de la commission sur ces deux amendements de suppression, monsieur le rapporteur indéfinie de l'emploi public puisse être considérée comme l'outil principal ou voir un outil incontournable de d'une politique publique, tenant compte du fait que on a évidemment un certain nombre de difficultés préma résoudre, souvent d'ailleurs plus en proximité, en lien avec les collectivités locales pour répondre aux besoins, aux attentes de nos concitoyens, il y aura besoin à par. De davantage d'effectifs de personnel et dans d'autres cas, une organisation différente y compris des services publics peut donner. peut donner. Davantage satisfaction en étant organisé autrement, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que par un espèce d'effet de sédimentation il ne faille jamais se remettre en question, c'est vrai, évidemment, des services publics de l'accueil des services au public qui sont concernées par vos amendements donc 2 avis défavorable. Monsieur le Ministre. Oui merci monsieur le président, madame la sénatrice brûlant, c'est vrai qu'il y a un changement par rapport à la précédente loi de programmation des finances publiques que l'objectif fixé pour les 5 ans qui viennent, c'est la stabilité de l'emploi public, ce qui ne veut pas dire effectivement que tout est figé puisque nous avons d'ores et déjà annoncé des créations d'emplois importantes notamment dans le secteur régalien, puisque nous avons annoncé 8500 postes de magistrats et personnels de justice supplémentaires dans les 5 ans qui viennent, pour poursuivre le réarmement du ministère de la justice, ça va aussi avec une augmentation budgétaire massivement déjà plus 40 % de budget pour le ministère de la justice, ces 5 dernières années on a annoncé 8500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, dont 3000 dès l'année prochaine vexé de ministère, on est déjà 17000 créations d'emplois dans la fonction publique, ce qui veut dire effectivement qu'il y aura des suppressions dans d'autres ministères et c'est le ministre du Budget, c'est-à-dire le principal pourvoyeur ces dernières années de suppressions de postes dans la fonction publique d'État, qui vous parle, c'est d'ailleurs un énorme un énorme effort qui a été fait par Bercy, mais qui était aussi le fruit de modernisation de l'apport du numérique, de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de la suppression de certains impôts comme la taxe d'habitation, maintenant la contribution à l'audiovisuel public qui a permis de faire ces redéploiements, donc il y aura des évolutions puisqu'il y a des créations mais au global sur le quinquennat effectivement nous souhaitons avoir une stabilité des effectifs publics en revanche ce qui me surprend un peu plus, c'est que, par cohérence avec le la trajectoire qui a été adopté par la majorité sénatoriale, c'est vrai que je m'attendais à ce qui est peut-être un amendement pour prévoir des suppressions de postes dans la fonction publique, puisque avec 37 milliards d'économies supplémentaires votés dans le cas des amendements qui ont été adoptées pour faire pour faire seulement un quart pour faire seulement un quart des économies supplémentaires qui ont été adoptées 37 milliards un quart seulement il faudrait supprimer 200000 postes de fonctionnaires. que la clé de répartition générale c'est que 10000 postes de fonctionnaires, c'est 500 millions d'euros, donc voilà c'était pour simplement pour insister sur cet enjeu de cohérence. Entendu, donc Monsieur. Oui, simplement, d'abord pour dire que dans le texte concernant la stabilisation des effectifs dans le texte du gouvernement il déprécié stabilisation nous avons-nous adopter un amendement pour considérer que c'était, c'était un plafond. Ce qui veut dire que dans l'objectif, monsieur le Ministre, on entend bien qu'il serait utile et qu'il faut penser à une réduction des effectifs, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on a un certain nombre de tous les ministères doivent être quelque part sur la ressource humaine analyser pour regarder avec des moyens nouveaux, parfois ce sont des moyens où il faut actualiser les capacités des équipes à travailler avec évidemment évidemment des moyens modernes qui permettent de gagner du temps, moi j'ai vu des choses assez intéressantes d'ailleurs dans une mission de contrôle enfin une mission plutôt sur la fraude, le contrôle de la fraude dont on voit qu'il y a des moyens très importants d'ailleurs dans ce cas-là, parce que ça produit des effets, on a même demandé des effectifs par redéploiement sur les 5 années qui viennent, mais il faut dire les choses, enfin je j'ai l'occasion de le dire, en commission, le ministère de l'éducation et le mieux doté de France, on a moins d'élèves, de, de, d'enseignants et on est quasiment en queue de peloton dans les enquêtes d'évaluation Pisa est-ce que c'est un gros mot. Et ce qu'il ne faut pas poser le la question et regarder de quelle manière on se développe et on répartit les effectifs ben pour moi c'est pas un gros mot et on aura l'occasion de le revoir dans les effectifs de la fonction publique, qui sont très nombreux : 150000 départs par an 30 % seulement pour la retraite, c'est aussi le travail de l'exécutif, c'est votre responsabilité, monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix, ces 2 amendements de suppression de numéro 5 et le numéro pardon 31, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Merci, abstention, ils sont pas adoptés, nous avons ensuite 2 autres amendements en discussion commune les numéros 18 et 54 Monsieur Bruillet présente le

vous avez évoqué les 8500 postes de justice ou ceux de la police, l'État et ses opérateurs auront aussi besoin de recruter des agents par exemple à météo France, face aux événements climatiques à l'Office national des forêts, qui connaît actuellement un mouvement social parce qu'on leur demande d'équilibrer leur budget par la vente, mais qui n'ont plus les moyens de la gestion de la forêt et alors qu'on vient de vivre des incendies dramatiques, il sera aussi nécessaire d'augmenter les services instructeurs des projets d'énergie renouvelable, au moins 100 selon France Énergie éolienne pour atteint atteint les objectifs que la loi sur l'accélération des ENR nous donnera, nous l'espérons du moins puisqu'elle viendra en discussion demain matin, il faut aussi être capable d'être réactif en terme de ressources humaines pour répondre à à ses besoins et d'ailleurs le gouvernement le sait bien puisqu'il a augmenté malgré tout 174 millions d'euros, soit 4,3 pour 100 les moyens humains de la structure gouvernementale, c'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement modéré pour une évolution raisonnée des schémas d'emplois qui laisse de toute façon au Parlement la main au moment des votes budgétaires mais qui indique très clairement que ça n'est pas en supprimant des postes qu'on est capable non plus de répondre à l'ensemble des besoins qui se font jour au vu des aléas et des crises qui se multiplient. Messieurs kaput pour l'autre amendement en discussion commune le numéro

nous ne pensons pas que nous pourrons atteindre la réduction de notre déficit telle que nous le demandons en ne tout en maintenant la stabilité des emplois sur le quinquennat donc l'amendement que nous et, en cela, nous sommes cohérents avec ce que dit le ministre, le ministre a raison, on peut pas demander la réduction du déficit tout en ne proposant pas tout en ne se fixant pas des objectifs ambitieux de réduction de la dépense, donc l'amendement qui vous est proposé propose sur le quinquennat de baisser le le le nombre d'emplois de 5 % % ça correspond peu ou prou à l'engagement du président Macron en 2017 d'une suppression de 120000 postes, j'ai bien compris que ça n'était plus l'engagement du dernier de de la dernière campagne, j'ai bien compris que ça n'était pas la proposition actuelle du gouvernement, la difficulté et pour les indépendants, nous ne voyons pas comment en cohérence, nous pourrons atteindre la réduction de notre déficit s'il ne nous ne nous fixons pas un objectif ambitieux de réduction de la dépense publique, c'est la raison de cet amendement. Alors il faut l'avis de la commission sur les deux amendements et ensuite on choisira. Alors ce sera pas le même avis sur les deux amendements, on va les prendre dans l'ordre sur le dix-huit du sénateur, c'est une demande de retrait, j'avoue qu'il faut, je me suis dit est-ce qu'il y a de la sémantique parce que je connaissais l'agriculture raisonnée ont l'évolution raisonnée des employes de l'État en fonction des besoins, je l'interprète en me disant que si les besoins sont réévaluée annuellement, sous-entendu : on a des besoins supplémentaires, le raisonnement c'est toujours à la hausse, vous avez compris qu'elle était parce que pour moi, raisonner, ça peut être aussi et bien sûr à la baisse, sinon le dit, on a un plancher, c'est jamais en dessous donc une demande de retrait sur l'amendement qui a été défendu à l'instant par le sénateur kaput je rends un avis de sagesse parce qu'effectivement cette question Monsieur le Ministre, vous avez l'occasion de dire on attendait vous avez une proposition qui s'inscrit dans le droit fil des propos d'un président de la République, élu en 2017 et réélu cette fois-ci, alors il a pas tenu sa promesse de 2017 mais peut tenir un engagement qu'il n'a pas pris, mais qu'il honorerait de réduire dans les capacités évidemment de chaque ministère, les effectifs, je le redis, 30 % seulement des 150000 emplois publics qui sortent chaque année. C'est pour la retraite, sur le reste, vous avez des capacités à renouveler et donc à trouver la juste proportion des choses très honnêtement, je pense que je vous le disais, il y a quelques instants, c'est, c'est un choix, mais c'est surtout aussi votre responsabilité puisqu'il faudra aussi que vous mettiez des moyens et vous soyez en cohérence avec les actions que vous préconisez. Monsieur le Ministre votre appréciation sur les deux amendements. défends au nom du gouvernement, la stabilité de l'emploi public, pour les 5 ans qui viennent, c'est vrai qu'il y avait, je le disais tout à l'heure un engagement pris par le candidat en 2017, le candidat Macron en 2017 avec un objectif chiffré de réduction de postes de fonctionnaires et ça n'est pas, qui n'a pas tenu. Mon engagement, c'est qu'il a assumé de revenir sur son engagement, il a dit, après la crise des gilets jaunes, qui était quand même marqué ce n'est pas le seul mot d'or de la crise des gilets jaunes, il y avait évidemment un enjeu très fort autour de la rémunération du travail mais il y avait aussi un enjeu sur la présence des services publics dans les territoires et on sait que la présence des services publics dans les territoires, elle passe aussi par des fonctionnaires qui sont au contact de nos concitoyens pour les accompagner dans leurs démarches être présent alors alors. Contact et donc on a assumé effectivement de sortir de cet objectif chiffré, mais quand c'est possible et quand ces produits par des réformes de structure effectivement pouvoir redéployer un certain nombre de postes et je le disais tout à l'heure, on prévoit de créer 8500 postes dans la justice 8500 postes dans la police et la gendarmerie, 3000 postes pour nos armées et c'est dans l'attente, en plus de la future loi de programmation militaire qui va probablement sur les dernières années, les quinquennat prévoir un certain nombre de créations de postes également donc ces créations de postes, rien que pour ça j'ai ça fait déjà 20000 postes de création, elles vont être gagées par des suppressions de postes dans d'autres ministres dans d'autres ministères, donc il y a déjà un effort qui est fait, j'imagine, monsieur le sénateur, qui a pu que à travers l'amendement que vous proposez, il y a d'abord l'enjeu de mettre dans le débat, cette question de l'emploi public et je pense que c'est toujours sans d'avoir ce débat, mais j'imagine que vous ne souhaitez pas ou vous ne visait pas baisser de 5 % les postes dans la justice, ni dans la police et la gendarmerie, ni dans les armées, et donc ça laisse un certain nombre de possibilités, monsieur le rapporteur général, je ne vous interpelle pas quand vous prenez la parole, donc moi la question que je pose est simple, c'est à ce moment-là, ou est-ce que vous les prenez les 125000 postes de fonctionnaires puisque c'est ça 5 % dans quel ministère est-ce ce que vous voulez supprimer, on a eu ce débat pendant la campagne présidentielle puisqu'une candidate à Madame Pécresse proposait de supprimer, je crois que c'était aussi 120000 ou 150000 postes de fonctionnaires et pendant toute la campagne présidentielle, on avait cette question mais finalement ou est-ce que vous voulez supprimer dans quel ministère dans quel administration on n'a jamais eu la réponse, mais encore une fois parce que c'est compliqué parce que nos concitoyens, ils nous demandent plus de service public, ou mieux de services publics sur un certain nombre de de de mission, nous on pense qu'on peut faire mieux avec une stabilité de l'emploi public en créant des postes pour la sécurité des Français pour la justice, pour nos armées et que ça veut dire qu'on va devoir supprimer des postes ailleurs mais dire qu'on va supprimer 125000 postes de fonctionnaires, sans préciser où est-ce qu'on les prend encore une fois, ça me semble pas justifier pas crédible, donc c'est une demande de retrait sinon avis défavorable.

je veux juste rappeler que on verra ça a sans doute en 2ème partie du PLF en tout cas je l'espère, mais cette année, il y a un petit changement, et il y a plutôt une évolution qui va dans le sens que vous appelez puisqu'on verra en 2ème partie que il y a six effectif et qui entend plein supplémentaires, vous voyez, donc ça peut quand même se faire parfois par des jeux de compensation et il arrive que, y compris le Sénat et la commission des finances écoutez parce que j'avais présenté un rapport sur ce thème, l'année dernière, juste qu'on garde ce point là, à l'esprit quand même, il peut arriver qu'on y arrive. Donc, nous pouvons voter maintenant sur l'amendement dix-huit de Monsieur, pardon monsieur Savoldelli vous souhaitez aussi expliquer votre. Oui la la, c'est quand même un moment important puisque. On joue 125000 emplois et en plus, les choses ont été dites. J'ai regardé, c'est juste un il y a un million neuf employes qui concerne l'état 489000 par ces opérateurs.

Et là, vous avez un problème, c'est que le ministre-qui vient de vous répondre, a aussi la sincérité de aussi de son côté, de dire ce qu'il fait. Donc moi j'ai regardé, il a raison, loi de programmation militaire, c'est à peu près 6000 emplois, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur 8500 policiers et gendarmes. Loi de programmation de la recherche et l'enseignement, ça nous fait à peu près 100200 recrutements. Donc ça fait 19700 les 20000 allez on ne va pas mais où ça se passe là. On est en train de supprimer la moitié des emplois publics dans des domaines. Si on écoute cet amendement. Donc il ne faut pas se raconter d'histoires, il y a une cohérence, il y a une logique, il y a un projet si c'est ce si c'est le vote Monsieur le Ministre, c'est un autre problème. Mais c'est quoi, moi je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'on va supprimer un moment des emplois par exemple dans l'enseignement et la recherche pour que ces emplois qui étaient publiques, deviennent des emplois privés parce que la demande avec la le besoin, il va être exprimée. Donc c'est un amendement extrêmement grave à mon avis pour nos notre cohésion et en même temps, qui porte un nouveau projet de société, celui de privatiser tout ce qu'qui a de la valeur ajoutée, voilà c'est tout, si ça vous va ça vous va ça, c'est un projet de société qui opposable suivant le point de vue qu'on a, c'est en gros suivant, c'est que moi, je pense, et nous pensons qu'il y a une série de service rendu à nos concitoyens qui relève vraiment du secteur marchand et qui n'a pas place dans le secteur public, par contre, il y a d'autres services rendus à la population qui ne doivent relever que du service public, là on est en train de toucher avec cet amendement, là en gros diminuer près de la moitié des emplois publics dans des, dans des domaines. Moi, j'irai pas régalien. Mais essentielle. c'est c'est un vote important et moi je pense que ça serait bien qu'on a un scrutin public tiens pour la peine. Monsieur Breuiller veut prolonger le débat quelles seront les 125000 emplois qui seraient supprimés, je me permets de lui retourner la question pour les 25000 puisqu'il y a à peu près dans les lois de programmation 25000 emplois nouveaux programmé donc quelles sont les 25000 qui seront supprimés dans les autres services publics d'État. Ensuite, madame-t-elle. Merci monsieur le président, ce débat est effectivement intéressant et moi je me méfie toujours des effets d'annonce, surtout quand ils sont quantitatif ce la quantité répond aussi un objectif de qualité et je pense qu'il faut qu'on soit effectivement vigilant, moi je ne partage pas tout à fait ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure parce que les employes ne sont pas forcément privés mais parfois il y a eu des transferts de fonction vers les collectivités, je prends l'exemple de l'urbanisme, je prends l'exemple de titres d'état civil qui précédemment été gérés par l'État et ont été transférés aux collectivités qui ont dû créer des emplois, donc je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur des annonces de suppressions d'emplois, par contre, Monsieur le Ministre, moi ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait une évaluation de l'ajustement des effectifs aux objectifs et aux évolutions de l'organisation, ce que je pense que dans notre pays, on a toujours tendance à entériner ce qui existe, par contre, vous le dites vous-même, on a aujourd'hui des besoins supplémentaires en matière de sécurité alors qu'un moment, on pensait que les besoins à les diminuer, donc la société bouge nos besoins aussi et je pense qu'il faut que l'État procède à des évaluations de ses services de fonction publique et l'évaluation, elle est largement qualitatif et on aura une meilleure adéquation des moyens et des besoins et du service à rendre. Que la ensuite.

avant vous aviez des directions départementales de l'équipement, vous aviez des directions départementales de l'agriculture et de la forêt bon tout été regroupés maintenant vous aviez quand même des services de l'État qui aider les élus de proximité, en particulier dans les petites communes pour faire des devis autrement maintenant quand on est maire de petites communes, ben, on se retrouve relativement, il faut le dire isolée, il y avait les services de l'État qui aidaient quand même largement maintenant ben tout a évolué, alors Monsieur le Ministre ou indiquer qu'il y a des des créations d'emplois à venir, notamment en matière de sécurité intérieure, je crois que c'est, c'est aussi une priorité, les gendarmes, les policiers mais pour former un gendarme ou un policier, il faut aussi du temps de l'autre côté il y a les transferts qui ont été faits depuis quand même pas mal d'années non plus en direction des autres la fonction publique territoriale, bon il y a quand même les polices municipales maintenant aussi compris il y a, il y a quand même des transferts, il y a les communautés d'agglomérations, communautés de communes compris aussi un certain nombre de compétences, le le problème des emplois, fonction publique d'état fonction publique territoriale et font fonction publique hospitalière, faut dire que réellement on est pour les les moyens humains, il convient d'avoir les moyens humains, c'est, c'est important, mais c'est vrai que c'est c'est un, c'est un problème important qui mérite réellement d'être souligné, je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous souhaitiez intervenir, je pense qu'ensuite on peut passer au vote, puisque le temps avance. Absolument, mais je pense qu'on ira plus vite sur d'autres parties du texte c'est un c'est quand même un élément fondamental quand on parle de notre fonction publique, on parle de notre État du sens qu'on lui donne des priorités qu'on lui assigne et de la manière dont on a à répondre aux problématiques qui se posent tous les jours dans la vie quotidienne des Français, ça mérite quand même d'avoir ce débat qui est un débat majeur et je pense que si on essaye de synthétiser tout ce qui se dit, c'est que on est tous d'accord pour dire que notre fonction publique telle qu'elle est telle que les effectifs sont répartis entre les différentes administrations n'a pas à être immuable pour reprend les propos de Madame Gatel, les besoins des Français évolue la société bouge, il doit aussi y avoir des évolutions, il y a aussi des priorités politiques qu'on se donne et c'est vrai que s'agissant de la sécurité oui on veut doubler le temps de présence de nos forces de l'Ordre sur la voie publique à horizon 2030, on veut créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires fléché, notamment dans les zones rurales et dans les villes moyennes, ça demande des effectifs supplémentaires, en l'occurrence 8 1500 postes sur le quinquennat trois mille dès la dès l'an prochain, on veut continuer à réarmer le ministère de la justice pour qu'il puisse traiter plus rapidement sanctionner plus rapidement aussi, ce qui est commis, ça demande des créations de postes, 8500 postes pour les magistrats, les greffiers, on veut continuer à renforcer nos armées, c'est au moins 3000 postes, donc on sait qu'il y a ces besoins-là moi ce que je dis, c'est que ce que nous défendons, gouvernement, ça me semble être une position équilibrée, c'est la stabilité de l'emploi public sur le quinquennat et donc ses efforts qu'il faudra faire dans d'autres ministères, j'ai été interrogé pour me dire : mais où finalement est-ce que vous pensez pouvoir faire ses efforts, je pense qu'il y a des ministères dans lesquels on continue à faire des réformes de modernisation qui permettent ensuite ben de redéployer un certain nombre d'effectifs et l'exemple de Bercy est un bon exemple : on a fait le prélèvement à la source, ça a permis d'alléger un certain nombre de postes qui était dédiée au recouvrement de l'impôt, on supprime la taxe d'habitation, la contribution à l'audiovisuel public, là aussi, ça permet d'alléger un certain nombre de fonctions, on développe de plus en plus le recours à l'Intelligence artificielle pour les contrôles fiscaux, plus de 50 % de nos contrôles fixes fiscaux sont aujourd'hui orientés par l'Intelligence artificielle, forcément ça libère aussi un certain nombre d'effectif, donc vous avez des ministères dans lesquels une modernisation, une numérisation permet de dégager des marges, je pense qu'il y a aussi du fait de la poursuite de l'amélioration de l'emploi dans notre pays et l'atteinte, on l'espère tous et on y travaille, c'est pour ça qu'on fait des réformes du plein emploi à horizon 2027 dans un certain nombre d'opérateurs et notamment Pôle emploi ça peut s'accompagner, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans les conventions de Pôle emploi quand vous avez la réduction d'un nombre donné de chômeurs : vous avez, avec une réduction d'effectifs qui est chiffré, ça peut aussi permettre de faire un effort, il y a des ministères dans lesquels on sait que les créations de postes nécessaires vont être moins importants ont donné tout à l'heure, l'exemple du ministère de l'éducation nationale, il y a 5 il y aura 500000 élèves de moins dans l'enseignement scolaire, dans les 5 années qui viennent, ça veut dire que pour garder un même taux d'encadrement auprès de nos élèves, vous aurez besoin de moins de créations de postes, voilà mais tout ça permet de gager entre guillemets les 20 ou 25000 créations qui sont prévus sur le quinquennat pour le domaine régalien, pour les 125000 suppressions qui sont proposés par l'amendement avec la baisse de 5 % là j'avoue que je vois mal aujourd'hui comment est-ce qu'on fait 125000 suppressions de postes, sans que ça touche à l'accès aux services publics dans nos territoires, pour les Français, c'est pour ça que vraiment demande de retrait ou avis défavorable aussi sur cet amendement. Je mets aux voix l'amendement dix-huit de Monsieur, avec avis défavorable de la commission également du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour.

la ville la commission et sagesse, l'avis du Gouvernement est défavorable, il est va être proposé ce procédé pardon au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Donc. Nous votons ainsi sur l'article 10 dans son ensemble. Qui est pour. Qui est contre. ne peut recompter, qui est pour. Qui est contre.

Merci monsieur le président, commettrions une erreur, c'est-à-dire de mettre beaucoup trop de rigidité dans les plafonds d'emplois des opérateurs de l'État, les opérateurs de l'État, je crois qu'il y en a plus de 400 on en a cité de tout à l'heure, météo France et l'Office national des forêts, leur situation sont extrêmement différentes, leur mission extrêmement différentes et là, en faisant en diminuant le plafond d'emplois à chaque fois qu'il y aura des vacances d'emplois y compris tout à fait involontaire dû à des difficultés de recrutement par exemple et ça peut arriver, il y a notamment des opérateurs de de l'État qui agissent dans le domaine de l'enseignement, on sait les difficultés de recrutement, aujourd'hui je pense qu'on a introduit une rigidité à la baisse, mais qu'on pourra regretter le jour où on aura besoin de pouvoir faire des exceptions et donc cet amendement est un amendement de suppression, pour ne pas infliger une règle trop rigoureuse. vie de retrait pardon. Ministre ma vie. Ils ne sont pas retirés. Une fois, 2 fois non donc je mets aux voix les trois amendements de suppression qui est pour. Qui est contre. Et ils ne sont pas adoptés donc l'article onze peut être mis aux voix qui est pour.

Merci monsieur le président, donc, cet amendement visa contester le le schéma des crédits par mission budgétaire proposée par le le gouvernement si indubitablement un effort et effet hein sur la le régalien cette trajectoire budgétaire contrainte en particulier par les les renoncements du gouvernement en matière de de recettes fiscales et je ne reviendrai pas ou aux amendements qu'on a défendu tout à l'heure, mais quand même, n'est pas à la hauteur, donc des un des enjeux que que connaît notre pays et qui nécessite un interventionnisme fort des pouvoirs publics, tennis, telle n'est pas le cas malheureusement dans le présent article. même avis les crédits prévus ne nous donne pas les moyens de répondre aux défis qui s'annoncent, notamment en matière de transition écologique vous fixer des niveaux de crédit sans connaître le niveau de recettes ni la conjoncture économique ni les situations critiques auxquelles nous devrons faire face, c'est la raison pour laquelle, nous vous proposons de changer d'indicateurs et de repères, de ne plus répondre à une crise par des coups de boutoir mais de préparer la résilience de la France, nous ne voterons non pas cet article qui ne pensent pas l'avenir de façon juste socialement, écologiquement et plus soutenable budgétairement.

effectivement, là on est sur un article qui consacrent les moyens dévolus à différentes missions budgétaires jusqu'en 2025 avec une pluri-annualité qui permet de connaître les intentions gouvernementales pour 3 ans, mais une trajectoire qui est là encore durci par la droite sénatoriale et là encore, comme sur le débat précédent qui concerne qui concernait l'emploi public, on aimerait bien avoir des précisions sur cette trajectoire durcit et ne pas en rester sur seulement à des mots du Style une trajectoire plus rigoureuse et ambitieuse dans la ligne d'un redressement des comptes publics et cetera, je pense que nos concitoyens aimeraient bien savoir ce qui se trame derrière, par exemple, on assiste là à la diminution de crédits pour 6 missions dont celle des relations avec les collectivités territoriales, elles apprécieront elles apprécieront d'autant qu'il a été rappelé à juste titre, tout à l'heure que un certain nombre d'emplois leur et leur ont été transférés au-delà de ces diminutions de moyens pour ces missions, il y a aussi la situation liée à l'inflation, c'est-à-dire des crédits qui font, qui vont s'éroder de fête du fait d'une inflation qui est largement sous- estimé, y compris lorsqu'on prend les données même du rapporteur, je ne citerai que les crédits par exemple de l'enseignement supérieur qui évoluerait de 9 83 % ça paraît pas mal comme ça, mais lorsqu'on regarde quels sont les les prévisions en matière d'inflation, on s'aperçoit que c'est 9 83 pour 100 fondent comme neige au soleil alors qu'il s'agit précisément puisqu'il s'agit de l'enseignement supérieur d'un investissement pour l'avenir de notre pays. Sur le principe de vouloir supprimer l'article et donc de supprimer toute trajectoire clairement mon point de vue, c'est pas un bon signal, je pense qu'on a besoin, je le redis de baisser la dépense publique, je le dis d'autant plus. Je dirais aisément que je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, ça fait 3 ans que la dépense publique augmente considérablement donc refuser de regarder les choses et de fixer une trajectoire à des réductions ne me paraît pas souhaitable et donc un avis défavorable pour les trois amendements amendements 7 20 et 33. Monsieur le ministre est l'avis du gouvernement. Avis défavorable pour les mêmes raisons. Je mets aux voix les trois amendements de suppression

Alors, très honnêtement, madame la sénatrice, je veux vous donner quelques explications parce que je peux pas me satisfaire d'une simple substitution du terme Euro constant en termes courant je veux vous signaler que ça signifierait une augmentation de presque 10 % supplémentaire de crédits de toutes les missions du budget général en 2025, hors pensions et donc, à défaut de recettes nouvelles, cela entraînerait un accroissement du déficit de l'ordre de 40 milliards d'euros, un avis défavorable. J'ai Ministre même avis. Je me vois cet amendement 45 faisant l'objet d'un double avis défavorable qui est pour. Contre. Abstention : il n'est pas adopté 2 amendements en discussion commune 46 de monsieur Savoldelli madame brûle, Il s'agit de majorer de manière conséquente les crédits dédiés à la mission Écologie développement et mobilités durables 9 milliards d'euros chaque année pour développer un effort extrêmement conséquent en matière de rénovation énergétique, je ne vais pas développer sur la crise que nous vivons aujourd'hui, qui nécessite de très gros investissements mais qui sont les économies de demain et il nous semble que dans les trajectoires à travailler il y a, particulièrement celle-ci.

très en décalage avec les discours de madame la première ministre si elles augmentent facialement 2023 7 en trompe oeil puisque, en fait, elle baisse si on additionne PLF épais par ailleurs elle continue ensuite à avoir une une trajectoire descendante, ce qui est en contradiction absolue avec la nécessité de se donner les moyens de la transition pour une société plus résilientes et moins polluante, d'après les estimations, conduite par l'institut de l'économie pour le climat Alfonsi si il faudrait entre 13 et 30 milliards d'euros de plus en faveur du climat si nous ne faisons pas ses investissements, nous ne serons pas capables de faire face à l'augmentation prochaine de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles, ah la perturbation croissante des écosystèmes du climat et à la raréfaction des ressources naturelles, il s'agit donc là d'une dépense responsable et d'un investissement d'avenir investir dès aujourd'hui dans la rénovation thermique, ça a été évoqué ou dans la construction de digues dans le développement de procédés indépendant du pétrole dans la protection contre les inondations dans la gestion des forêts, c'est demain, ne pas avoir à payer pour pour réparer nos dégâts en fait, on ne veut plus rester dans des réponses au coup par coup aux crises nous voulons une politique résiliente qui décide d'investir fondamentalement en direction de cette mission Écologie développement et mobilités durables. Sur l'amendement 46 l'avis du rapporteur général. SNCF, réseau et du service public de l'énergie, il me paraît d'ailleurs difficilement applicable pour une raison assez simple, c'est qu'il prévoit une augmentation des la loi de finances pour 2022, donc de manière c'est ainsi rédigé rétroactif, ce qui ne me paraît pas possible. Et entre nous, s'il suffisait de modifier un chiffre dans un tableau pour faire d'une politique aussi importante et ambitieuse, une réalité, je pense que ça fait un certain temps qu'on aurait pu mettre ou inscrire des crédits supplémentaires, la question de la rénovation énergétique, je le dis d'autant plus librement que depuis des années, j'ai déploré le manque de moyens mis sur la rénovation énergétique parce que, et on l'a encore vu cette année, c'est beaucoup du mono geste c'est mal suivi c'est mal accompagnée, c'est donc de l'argent jeté par les fenêtre si j'ose dire.

si vous aviez regardé c'est une mobilisation de moyens publics et privés, et pour être tout à fait honnête je pense d'ailleurs que c'est pas le rôle de l'État à lui seul l'état, il doit évidemment impulser et donner un cadre d'action doit-il aller d'ailleurs jusqu'à, jusqu'à une planification parfois, je me pose la question parce qu'avant de planifier, il faut d'abord affirmé et faire partager une stratégie et ensuite l'État et l'ensemble des acteurs publics, essayer d'avoir un travail coordonné mais surtout et peut-être plus encore, je pense que les acteurs privés ont un rôle décisif, j'ai vu que la BCE faisait des remontrances, même plus que ça aux banques, moi je crois vraiment que la finance verte si elle est je dirais pousser jusqu'à la mise en oeuvre de manière concrète et au-delà de de d'un simplement d'un affichage un peu à l'image du budget Vert que le gouvernement a vanté pendant 2 ans, je pense que, à ce moment-là peut être ensemble on peut gagner la partie, et un avis défavorable, une demande de retrait sinon défavorable. Maintenant l'avis du gouvernement sur ces deux amendements. Même avis. Entendu donc de où nous allons voter sur l'amendement numéro 46 de monsieur Savoldelli avec double avis défavorable qui est pour. Bon. Qui est contre. Est pas adopté et ensuite sur l'amendement 21 de Monsieur Bruillet avec également double avis défavorable qui est pour. Qui est contre, n'est pas adopté non plus 2 jours sur cet article, nous avons l'amendement 58 bis et qui va être soutenu par monsieur

Il est défendu, il s'agit d'augmenter les crédits de la mission Travail, emploi et recherche et enseignement supérieur pour former suffisamment nos ingénieurs. Entendu monsieur rapporteur général. monsieur le sénateur qu'il suffise d'augmenter les moyens, sans chercher par ailleurs à regarder les économique qu'on modifiera peut être, j'allais dire substantiellement, mais surtout en profondeur les politiques donc attention aux augmentations de crédits non ciblées. non ciblées. J'. Défavorable. Entendu donc je mets aux voix l'amendement 58 bis de nos collègues indépendants avec le double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Et il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 12 maintenant, qui est pour.

mes chers collègues, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, à l'Assemblée nationale, le gouvernement intégrée au texte retenu au titre de la procédure 49 3, plusieurs amendements qui augmente les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour cette année, à savoir une majoration de la DGF à hauteur de 200 millions d'euros, ayant pour objectif, d'une part d'augmenter la DSU, ainsi que la dotation de solidarité rurale de 90 millions d'euros chacune entre 2000 22 et 2023 et d'autre part d'augmenter la dotation d'intercommunalité de 30 millions d'euros, premièrement, deuxièmement une majoration supplémentaire de 110 millions d'euros de la DSR pour renforcer le soutien apporté aux communes rurales, troisièmement, une progression de 30 millions du PSR de compensation des exonérations de fiscalité locale, c'est l'article 11 squatter qui supprime les conditions relatives à la cohabitation requises pour le bénéfice d'allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et enfin quatrièmement, la mise en place au titre de 2023 d'un nouveau filet de sécurité pour les collectivités territoriales, y compris, départements et régions face à la hausse des dépenses d'énergies pour un montant d'un milliard 5 ces dispositifs viennent mécaniquement augmenter le plafond des concours financiers de l'État, soit pour une seule année, c'est le filet de sécurité, soit de manière pérenne avec la majoration de la DGF et l'augmentation des exonérations de fiscalité locale, monsieur le Ministre, vous ne prévoyait pas d'amendement, tirant les conséquences de ces votes à l'Assemblée nationale sur le plafond, telle que définie à l'article 13 de cette loi de programmation des finances publiques, pouvez-vous nous en donner la raison et à quel moment de la procédure, comptez-vous procéder à cette modification que je qualifie d'indispensable.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer les plafonds des concours financiers à des stations, des collectivités locales proposées par le gouvernement et qui ne prennent pas en compte ce qu'qui a évoqué le rapporteur général précédemment, vous savez que les collectivités locales sont amenés à se substituer en matière de service public à l'État, qui s'est retirée des territoires au cours de ces dernières années, ce qui génère des charges particulières, on l'a vu en matière de d'implantation des francs service ou les collectivités assume à peu près 50 % des charges de ces nouveaux dispositifs concernant les les services publics, il y a des transferts de charges qui ne sont pas ou qui risquent de ne pas être complètement financiers on pense particulier aux routes nationales et puis il y a des besoins nouveaux qui émergent, bénéficiant notamment dans le domaine de la jeunesse, mais également, s'agissant des des personnes âgées, il faut rappeler que les collectivités locales génère 70 % de l'investissement public et que il y a devant nous des enjeux importants en matière de transition écologique à la fois au regard des ses activités propres des collectivités locales, mais également en matière d'accompagnement des acteurs économiques, publics comme privés, les plafonnement qui sont prévues aujourd'hui, conduirait à une évolution des recettes en volume inférieur à l'inflation, donc une perte de pouvoir d'achat, donc de marges de manoeuvre financières pour l'avenir et donc il est préférable, plutôt que de fixer des plafonds aujourd'hui et avec des échéances qui vont jusqu'en 2027 de laisser le soin au gouvernement et le parlement de définir en fonction des besoins qui émergeront en fonction des évaluations qui pourrait être plus précise de définir les plafonds nécessaires chaque année. Vous voyez par l'amendement 22. peut être un des plus puissants outils de réponse aux crises parce qu'il y a une agilité dans les collectivités territoriales, parce qu'il y a une diversité de politique portée par la diversité politique des élus qui dirigeait collectivités et c'est la raison pour laquelle à cet article qui, pour nous, consacrent l'austérité budgétaire imposée aux collectivités territoriales pour les 5 prochaines années, nous demandons la suppression de cet amendement, nous ne demandons pas que cet amendement la la suppression de cet article qui met pour nous des collectivités au pain sec et je voudrais dire, il appartient au législateur d'apprécier lors de l'examen de chaque projet de loi de finances, le bon niveau des dotations de soutien versée aux collectivités locales, au vu de la conjoncture économique des recettes des dépenses des circonstances et des initiatives prises par ces collectivités, voilà la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article et je confirme, Monsieur le Ministre, que vous ne m'avez pas convaincu, il n'y a pas de hausse des moyens lorsque cette évolution est inférieur à l'inflation. Et Madame brûle, hein, pour l'amendement trente-quatre. Merci, je crois en effet que cette loi de programmation est extrêmement grave pour les collectivités, alors on y viendra, mais ensemble nous allons supprimer l'article 23 que les associations d'élus qualifient d'un pacte de défiance et qui est une sorte de contrat de Cahors revisité, mais presque encore plus intrusif dans la libre administration des collectivités et avec les plafonnement qui sont proposées dans cet article, on retire, là aussi, des moyens importants aux collectivités puisqu'en N'Euro constant, cette baisse s'élèverait à plus de 4 milliards d'euros, je ne vais pas développer à l'heure qu'il est sur la situation que vivent aujourd'hui les collectivités face à l'augmentation des coûts de l'énergie face à l'augmentation du point d'indice, qui n'est que très très partiellement compensé face à l'augmentation des matériaux, alors qu'il y a des investissements, notamment en matière de transition énergétique a opéré, je n'évoque pas non plus les les denrées alimentaires et cette situation semble. Pour partie structurelle, en tout cas durable pour les années à venir, et donc il nous semble que ces plafonds sont une très très mauvaise trajectoire pour nos collectivités. Monsieur le rapporteur général sur les trois amendements de suppression. Ce sera 3 avis défavorable je confirme une fois de plus, qu'on a besoin d'avoir une trajectoire quinquennal, y compris pour les concours financiers apportés par l'État aux collectivités territoriales, je crois que cette trajectoire, elle ne doit pas être une une contrainte. Qu'elle doit pas être contraintes pardon par des évolutions dynamiques d'ailleurs de certains concours qui viendrait diminuer les les PSR ou les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, c'est d'ailleurs dans cet objectif que j'ai proposé un amendement qui vise à sortir la TVA affectée aux régions de l'enveloppe normée c'est-à-dire strictement plafonné des concours financiers la TVA des régions coup tout comme le FCTVA pourra connaître une évolution dynamique même au-delà des montants prévus à l'article 13 sans que ça Vienne, diminuer les autres concours par ailleurs, je note que cette trajectoire est également en hausse de 1 milliard 4 et que cette hausse concerne aussi bien le FCTVA que la TVA aux régions et les autres concours financiers. Oui, merci Monsieur le Président, je pense que ce serait une mauvaise idée de supprimer cet article. Parce qu'on prévoit une programmation des finances publiques sur 5 ans, c'est plutôt protecteur pour les collectivités locales que dans cette programmation, il y a une trajectoire sur les concours financiers de l'État. Parce que c'est aussi une garantie pour elle. Et si on met pas de trajectoire, le risque, surtout dans un contexte où on nous demande de faire beaucoup d'économies supplémentaires qu'il n'y a pas de garantie pour les collectivités locales du maintien des concours financiers bah, le risque c'est que c'est là qu'on avait trouvé des économies, donc c'est aussi une garantie pour elle, pour ne pas revivre à ce qu'elles ont vécu au moment du quinquennat 2012, 2017 avec des baisses massives de DGF voilà, là au moins les choses sont sont garantis, c'est important ce que vous voyez comme un plafond, moi je le vois surtout comme aussi un plancher, puisque c'est ce qui garantit que leurs concours financiers ne vont pas baisser, ils vont même augmenter pour répondre au rapporteur général où il y aura une coordination à faire, notamment avec la revalorisation de DGF de 320 millions d'euros, qui a été annoncé par la première ministre classiquement dans Des LPFP la coordination se fait plutôt en toute fin de navette en toute fin de texte pour tenir compte de ce qui s'est passé dans les textes budgétaires mais il y aura cette coordination à faire sur le filet de sécurité, comme c'est un dispositif temporaire sur 2023 ça sera intégré mais c'est temporaire sur 2023 c'est pas sur l'ensemble de la programmation, moi ce que je veux rappeler, quand même, c'est qu'avec la trajectoire qui est prévu, c'est 31 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour les collectivités locales de 2022 à 2027, je le dis parce que parfois dans les débats, on a l'impression que les dépenses des collectivités locales vont baisser, non elle ne vont pas baisser, en tout cas ce qui est prévu, c'est important de se donner un cadre, on le fait pour l'État pour les collectivités locales aussi, ce qui est prévu, c'est que les dépenses progressent de 31 milliards d'euros de 2022 à 2027 ce qui va permettre évidemment une progression pour les dépenses de fonctionnement nécessaire mais aussi pour l'investissement dans les dernières prévisions qui sont faites par la direction générale du Trésor on prévoit une très forte augmentation de l'investissement des collectivités locales, dans les années à venir, si on compare 2 mandature a mandature, ce qui est prévu aujourd'hui par les prévisionnistes et les analystes, c'est que sur la mandature 2020, 2026 il y aura un investissement en hausse de 28,2 pour 100 par rapport à la mandature 2014, 2020 donc c'est évidemment très important, donc voilà ce qu'on souhaite, avec cet article, c'est évidemment conforter les collectivités locales, leur donner les moyens de continuer à agir et à investir, et je crois qu'on partage tous cet objectif, donc : avis défavorable. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Biya qui la parole.

il y a 200 ans de Napoléon disait qu'on ne gouverne bien de loin on administre bien que de prix il y a 40 ans ici, Gaston Deferre présenté la loi de décentralisation et depuis, on est au point mort, ne demande des crédits pour le travail et l'emploi, que je sache, la région a la compétence, les font faire les régions donnant aux régions les moyens d'agir, on a parlé de mobilité, les régions, la compétence transport les les régions agir mais non on a décentralisé, mais on a gardé la même au charme de finances au moins au niveau de l'État, alors moi je préconise, comme je l'ai eu dans ma DG. Que l'État donne les moyens, gros régalien et Dieu sait si la justice a besoin de moyens si la sécurité a besoin de moyens si la défense a besoin de moyens et le reste, ce qui n'est pas, régaliennes que dans le cadre de l'outil que le contrat de plan État-Région on ne donne les moyens aux collectivités qui en responsabilité prendre eurent par le dépense pour exécuter le reste. Monsieur Delcroix c'est demandé la parole est là. Merci monsieur le président, moi je voudrais interroger Monsieur le Ministre, sur un problème particulier aujourd'hui les collectivités perçoivent la CVAE c'est une ressource pour qui leur est propre pour environ 8 milliards d'euros, le gouvernement prévoit de supprimer la CVAE pour moitié presque en 2023 et l'autre moitié en 2024 qui sera remplacée par une une fraction de TVA qui devient donc une une un concours financier de l'État finalement cette fraction de TVA est-ce que cette donnée est intégré dans la programmation des concours financiers de l'État aux collectivités. Madame Gatel. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi, je ne doute pas du tout de vos explications que vous maîtrisez parfaitement toutefois néanmoins et cependant, on a vu des trajectoires explosé en plein vol, parfois et je pense que si nous avions aujourd'hui une loi de programmation pluriannuelle et que nous avions à faire face à nous adapter parce qu'il y a eu la crise sanitaire aujourd'hui il y a le problème de l'énergie qui va coûter 11 milliards d'euros supplémentaires en année pleine aux collectivités, plus l'inflation, monsieur le Ministre, moi je ne demande qu'à vous croire quand on dit que l'investissement des collectivités va augmenter en l'état actuel des choses, vous le savez très bien, il y a des collectivités qui font des Budgets d'investissement à zéro je salue l'amortisseur pour l'électricité que vous avez proposé parce qu'il est extrêmement simple, voilà par contre le bouclier la ministre, madame la première ministre, a dit l'autre jour, c'était très touffu et monsieur le maire, expliqué qu'il a pas fait Polytechnique, ce qui est mon cas, donc je pense que je ne comprends pas très bien le bouclier tarifaire qui part d'une bonne intention, mais je dis : Monsieur le Ministre, ce qu'on ait une loi programmation que l'on dise : voilà la trajectoire je suis OK mais il me semble, peut-être imprudente nous enfermer aujourd'hui dans des chiffres, je ne suis pas sûr qu'on les tienne et je pense que les collectivités sont responsables ne demande pas la charité à l'état, elle demande juste à pouvoir exercer convenablement les services au public que l'État leur a souvent délégué donc moi je vous avoue, c'est pas leur tardive qui me ferait commettre une erreur mais je voterai cet amendement comme un amendement d'appel.

Parce que je me disais on on va voter majoritairement pour les trois amendements précédents. Donc, je me disais : je vais le retirer mais obligé de le laisser parce que c'est un amendement de repli.

moins de 4 milliards entre 2016 et 2017 et là vous arrivez moins de du 9 milliards entre 2017 et 2018 quand je fais les comptes, ça fait plus de 13 milliards de DGF qu'ont été enlevés aux collectivités territoriales la preuve c'est que on peut affirmer une volonté après. Et vous en savez quelque chose comme comme ministre, j'ai regardé. 2018, 2021. Les concours financiers ont été supérieurs de 7 13 milliards en exécution. Par rapport au montant inscrit. Donc il y a plusieurs de mes collègues de sensibilités différentes qui viennent de s'exprimer. On ne peut pas corseté les choses de ça veut pas dire là. On ne peut pas les enfermer, de cette manière-là, parce que qu'est-ce qui se passe avec les collectivités territoriales, c'est qu'elles ont une capacité d'initiative, une capitale de réactivité une captivité de proximité à des besoins qui s'expriment. Et ça, ça on ne peut pas tout rentrer dans des cases dans des logiciels dans un encadrement. Donc et et et la preuve c'est que vous avez été obligé d'augmenter d'ailleurs. Donc à partir de là, cet amendement est un amendement de repli, c'est pour ça que le le mot, et là c'est pas une affaire de sémantique remplace courant par Constant parce que, au minimum, restons constants du point de vue des relations de confiance qui était ouais s'établir entre l'État et les collectivités territoriales sur la base de la libre administration. Voilà c'est c'est ce que nous soumettons à l'approbation de l'hémicycle. Monsieur le rapporteur général sur l'amendement 47. Alors, Monsieur le Sénateur, Savoldelli effectivement la hausse en euros courants d'un milliard Correspond en euros constants. à une baisse de 2 milliards 9 sur la période 2023 2027. Mais. il nous paraît important et nécessaire de trouver ce que j'appellerais un juste équilibre entre la protection des ressources de nos collectivités et une gestion rigoureuse de leurs finances. Plusieurs éléments, d'abord pour protéger, pour les protéger au mieux, on a modifié cet article pour que le dynamisme potentiel de la TVA affectée aux régions ne viennent pas affecté ni contraindre les autres concours financiers, raison pour laquelle on la sortie de l'enveloppe normée, deuxièmement le la suppression de l'article 23 de l'aile, PFP donne ou redonne de la liberté aux collectivités sur leurs dépenses de fonctionnement, enfin 3ème élément, on travaille dans le cadre du PLF sur un nouveau filet de sécurité pour 2023, de manière à compenser. Tout ou partie de la hausse, notamment des dépenses énergétiques des collectivités et je pense qu'avec ce dispositif. On répond suffisamment aux préoccupations des collectivités mais je crois aussi que nous devons. Montrer que les collectivités ne s'exonère pas l'État, encore moins d'où la trajectoire que nous proposons d'une partie d'effort à faire pour redresser la situation et réduit et c'est commencer à réduire le niveau de notre endettement. L'avis du gouvernement. Même avis pour les mêmes raisons. Très bien, donc je mets aux voix l'article l'amendement 47 présenté par Monsieur Savoldelli avec double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Y a-t-il des abstentions et ne pas adopté à titre documentaire, mes chers collègues, nous avons franchi la moitié du nombre des amendements en discussion et ça nous a pris une donc il est pas très difficile de prévoir la suite nous passons à 3 amendements en discussion commune. Nous commençons par le, 55 présenté par monsieur Très rapidement, monsieur le président, c'est un amendement qui est en cohérence avec l'amendement que j'avais déposé à l'article 9 qui vise à limiter à 1 % par an les dépenses de l'État, donc cet amendement lui visait a affirmé que les collectivités contribuerait à la même hauteur que l'État et pas plus à la maîtrise des dépenses publiques à partir du moment où, sur l'insistance de la Commission, j'avais retiré tout à l'heure là l'amendement à l'article 9 je retire également celui-ci.

je propose d'inscrire dans la trajectoire de la programmation pluriannuelle des finances publiques, une évolution de de du fonds de compensation de TVA qui permettent de tenir compte de la situation actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui reste des collectivités qui bénéficient de la TVA, l'année même de l'investissement, d'autres l'année en Inde, plus celle qui avait participé au plan de relance en 2008 et puis les autres collectivités s'entraînent plus de, or la plupart des actions des actions sont menées aujourd'hui de façon contemporaine, c'est-à-dire qu'on a par exemple l'imposition sur le revenu qui est contemporaine, on a aussi le versement d'un certain nombre de prestations qui est contemporain pourquoi conserve-t-on à remboursement aux collectivités territoriales de la TVA, 2 ans après l'investissement, cela n'a plus de sens, donc il importe de traiter cela dès à présent et je propose donc de faire cet effort de supprimer le plus de en 2023, comme ça il n'y aurait plus que pour les communes, un de plus, hein, l'idéal aurait été d'aller jusqu'à Rennes mais l'effort financier à souscrire serait trop important et de décalé sur la période, sur les 4 ans à venir, l'incidence budgétaire, ce qui fait que l'incidence en fait neutre, donc voilà le sens de cet amendement. Et l'amendement 67 du gouvernement. Oui, c'est un amendement qui rétablit la TVA des régions dans les. Concours financier de l'État, ça avait été supprimé en commission, je crois que ça avait été supprimé, monsieur le rapporteur général, parce que vous vouliez être sûr que ça ne rentrait pas dans l'enveloppe normée et que, au final, la TVA des régions, on allait du coup pas de peser sur les concours financiers aux autres collectivités locales, ça n'est pas le cas puisque la TVA des régions ne sera pas prise en compte, n'est pas pris en compte dans l'enveloppe dite normée pour autant la TVA des régions ex-DGF fait partie des concours financiers, c'est donc normal qu'elle soit mentionné dans le tableau, mais je le rappelle, je le redis, pour la clarté de tous, elle ne sera pas prise en compte dans l'enveloppe dite normée, donc il n'y a pas d'impact sur les concours financiers pour les autres collectivités locales. Très bien l'avis du rapporteur général sur les deux amendements. Alors sur le premier pour le sénateur Calvet, 2 éléments de réponse j'ai entendu parler d'une neutralité, je me dois quand même de donner le coût de la mesure telle qu'elle est proposée sur la seule année 2023, le coût serait de 5 milliards d'euros, à un moment où on demande de de maîtriser les dépenses, deuxièmement, cette réforme viendrait d'ailleurs percuté la réforme de l'automatisation qui s'applique cette année aux bénéficiaires du FCTVA en année N et qui s'applique en 2000 22 et 2000 23 au bénéficiaire ne plus hein et ne plus de raison pour laquelle j'émets un avis défavorable, monsieur le Ministre, le gouvernement et le Parlement 2018 ont souhaité remplacer la DGF des régions par une ressource dynamique, c'est donc à mon avis, pas pour la plafonner désormais et il ne me paraît pas envisageable que le dynamisme de cette TVA génère une baisse des autres PSR par ailleurs, et contrairement à ce qui était indiqué dans l'objet de l'amendement en 2017 lors de la précédente LPFP le texte déposé par le gouvernement prévoyait d'inclure dans le plafond, la TVA affectée aux régions, ainsi que le FCTVA et c'est d'ailleurs un amendement à l'Assemblée nationale qui avait permis de sortir la TVA affectée aux régions de l'enveloppe plafonnée des concours financiers, ce sera donc, là aussi, un avis défavorable. Je n'ai pas de demande d'explications de vote Monsieur Ministre ou les et je pense que nous aurons de beaux débats et de beaux moments dans le PLF sur la question du FCTVA on a déjà commencé, dès cet été, notamment à l'initiative de la sénatrice avare, très active sur ce sujet-là, à l'évidence, il faut faire un bilan et tirer des enseignements de la dernière réforme du FCTVA se poser toutes les questions sur l'assiette sur les années de référence mais c'est objectivement plus un débat de PLF qu'un débat de LPFP donc avis défavorable pour cette raison et vraiment je veux rassurer le rapporteur général sur la question de la TVA des régions quand une fois ses protecteurs pour elle que d'inscrire leur TVA dans la programmation des concours financiers sinon on met un peu en risque la stabilité budgétaire des régions, première chose et 2ème chose je le redis, ça ne rentre pas dans l'enveloppe normée vraiment donc il y a pas d'impact sur les concours financiers aux autres collectivités locales.

rien à voir avec le problème qui est soulevé le problème qui est soulevé, c'est qu'il existe 3 régimes de remboursement de TVA et de l'automatisation et simplement un logiciel qui permet de rendre automatique le versement mais ça ne

Qui est contre. Donc il est pas adopté l'amendement 67 du gouvernement avec avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il est pas adopté, non plus, je mets aux voix, l'article 13. Qui est pour,

Oui, c'est un amendement qui vise à rétablir attendez, excusez-moi, c'est un un amendement qui supprime toute référence. Aux dépenses dont l'impact est considérée comme mixte sur l'environnement, selon la classification du budget Vert de l'État en fait vous avez adopté en commission, une mesure qui vise à considérer que les dépenses considérées comme mixte dans le budget sont considérés comme défavorables pour l'environnement, or, par définition, si elles sont aujourd'hui mixte, c'est parce que elles peuvent avoir, par certains. En biais des. Impact favorable et par d'autres, un impact défavorable, je vous donne un exemple : pendant longtemps, les transports ferroviaires ont été considérées comme des dépenses, je crois qu'il y a une partie importante maintenant qui a été rebasculer en dépenses favorable mais vous avez encore dans les transports de personnes certains qui sont considérés comme mixte alors qu'on sait qu'ils ont pour une certaine partie un impact favorable sur l'environnement donc pour ces raisons-là, on souhaite maintenir la qualification et la classification telle qu'elle était présente dans le budget Vert. Il y a un ami du la commission sur cet amendement, monsieur le rapporteur général. En fait, il a, il y a 2 parties : la première, qui on va dire, est intéressante c'est-à-dire le l'objectif du ratio que défini cet article qui est de suivre finalement l'évolution respective des dépenses favorables et défavorables au climat, sachant que les dépenses mixtes n'apporte finalement qu'une information limitée et que leur montant d'ailleurs réduit, on pourrait donc envisager de retenir seulement le ratio des dépenses favorable et des dépenses favorables sans ajouter au numérateur ou au dénominateur les dépenses mixtes, par contre la la deuxième partie de l'amendement revient sur des avancées de notre travail en commission, ce que la diminution de 10 % du poids relatif des dépenses défavorables qui est prévu dans la version initiale du projet de loi nous paraît insuffisante et surtout qu'elle n'est pas réellement significative compte tenu du faible poids des dépenses côté par rapport à l'ensemble de budget, je souhaite que nous en restions la diminution de 20 pour 100, telle qu'elle a été adoptée en commission, d'où l'avis défavorable à cet amendement.

Et contre n'est pas adopté, donc nous votons sur l'article 14 qui est pour. Contre. Abstention : il est adopté. Article 15 un amendement 69 du gouvernement. Oui, c'est un amendement qui rétablit le bornage temporel et le dispositif d'évaluation pour les aides aux entreprises par d'autres entités que l'état il conserve l'ajout de la commission des finances du Sénat visant à l'établissement d'une liste. Au moins annuelle des dispositifs d'aide aux entreprises mais il supprime la référence à un arrêté ministériel pour l'établissement de ladite liste, je rappelle que c'est une mesure importante qui vise à borner les aides aux entreprises qui sont créés dans le temps, là je pense que ça devrait quand même satisfaire un certain nombre d'intervenants sur ce sujet-là. On propose désormais que toute aide aux entreprises soit bornés automatiquement dans le temps, c'est-à-dire qu'elle puisse pas aller au-delà de 5 ans c'est ça. Voilà 5 ans maximum, et que si on veut la prolonger ou la renouveler, ben il faut une évaluation, il faut que le Parlement décide souverainement de le faire, donc ça me semble être une mesure de bonne gestion, il y a eu un amendement adopté en commission des finances, qui visait. à restreindre aux seuls. Aide aux entreprises, instaurée par l'État, nous, on considère qu'il faut le faire pour l'ensemble des aides aux entreprises et donc on propose un rétablissement mais on tient compte de d'un certain nombre d'ajouts qui ont eu lieu en commission des finances que j'ai évoqué il y a un instant. Alors dans une partie de de l'amendement finalement vous introduisez enfin le gouvernement introduit une confusion et il revient sur une modification que nous avons apportées en commission effectivement qui précisé que l'Arctique se limiter aux dispositifs d'aide par l'État, c'est une modification que j'appellerais de bon sens, puisque l'article 15 qui fait partie de la section intitulée le cadre financier pluriannuel des administrations publiques central, il me paraît donc étrange qu'ils prétendent s'appliquer à des régimes d'être définie par d'autres autorités par exemple, les collectivités locales territoriales ou et et l'Union européenne, du coup, le périmètre de l'article devient particulièrement large et assurément mal défini et les conséquences juridiques d'un encadrement de ces régimes par l'état nécessiterait, à mon avis, d'être étudié de plus près et à ce stade, le gouvernement n'a apporté aucun élément sur la portée qu'il entend donner à cet article, d'où l'avis défavorable. Monsieur le Ministre. très rapidement, et pas rallonger mais il s'agit pas de dire que le sujet dans le périmètre, c'est les collectivités locales ou pas, les collectivités locales, on parle surtout des opérateurs en fait les opérateurs de l'État qui ne sont pas pris en compte dans la rédaction, que vous avez apporté un exemple l'ASP qui est destinataire d'un certain nombre de dispositifs du coup des dispositifs d'aide aux entreprises qui passent par l'AFP, ne serait pas pris en compte, moi j'entends comme c'est le gouvernement qui propose, mais, mais je veux dire c'est c'est objectivement de bonne gestion et on retient en plus on retient des ajouts qui ont été faits au niveau de la commission, on retient des ajouts qui ont été apportées par votre commission donc voilà mais évidemment. Monsieur rapporteur général. Non, le ministre a bien compris, j'entends ces explications s'il y a des améliorations apportées, elles feront l'objet de la navette considérer qu'ici, le Sénat et souverain. Je mets aux voix l'amendement 69 du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Permettez-moi de recompter, qui est pour.

ou l'extension d'aide aux entreprises, a une durée de 2 ans, et non pas 5 ans effectivement parce qu'il y a besoin d'évaluation et, si vous me le permettez, je trouve qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux en matière d'évaluation des aides publiques apportées aux entreprises et c'est à comparé à ce que vous suggérez que les collectivités face, c'est-à-dire que les collectivités, vous voulez les soumettre à une trajectoire extrêmement dur, un objectif de suivi de leurs dépenses de fonctionnement avec les moins 0 5 par rapport à l'inflation. Avec l'exclusion de subventions de l'État, si elle ne respecte pas ses trajectoires, on aimerait que le gouvernement et l'État soit aussi rigoureux vis-à-vis de l'aide accordée aux entreprises. nous, on propose de le borner à 3 ans pour la lignée notamment sur les dispositifs de niches fiscales et donc de passer de 5 à 3 ans. Et Monsieur kaput pour le groupe des Indépendants de 56. c'est comme tout à l'heure dans l'autre sens, je partage nous partageons évidemment l'objectif de bornage dans le temps, la difficulté technique, c'est qu'un bornage de 5 ans ça correspond pour une entreprise à des investissements de moyen terme, or, les entreprises ont besoin de stabilité, de visibilité et de sécurité juridique et fiscal, c'est la raison pour laquelle un délai de huit ans qui correspond à des investissements de long terme et techniquement plus pertinent.

c'est le l'objet du texte cette je pense s'agissant parce que je, je réponds également sur finalement une réflexion qui pourrait tendre à dire : on prend le la même durée que pour les dépenses fiscales, je crois quand même que, s'agissant des dispositifs d'aide aux entreprises, il faut souvent un peu de temps pour la diffusion et la connaissance donc deux ou trois ans me paraît un temps un peu trop court 8 ans assurément trop long donc demande de retrait sinon avis défavorable pour les trois amendements.

Contre, il n'est pas non plus adapté et le 56 et retiré, nous passons au vote sur l'article 15 lui-même qui est pour.

Merci monsieur le président, donc, comme vous le disiez, c'est un amendement de suppression de l'article 16 cet article qui vise à marquer un objectif indicatif d'évolution des dépenses locales alors certes, c'est un objectif indicatif, ça n'est pas le plus grave, à partir du moment où l'article 23 été en tout cas en commission supprimer ceci dit cet article indicatif, il montre bien une volonté d'une pression à la baisse alors le ministre dira que ça n'est pas à la baisse et pour en maîtriser l'augmentation des dépenses des collectivités locales, comme si elles étaient le problème comme si elle n'était pas souvent contraintes et notamment face à un certain nombre de crises que nous avons rencontrés que nous rencontrerons peut être nous pend et comme si, par ailleurs, enfin, ces chiffres ont été définis, sans tenir compte de la future inflation, ils n'ont pas du tout la même valeur, suivant l'inflation qui aura lieu dans la période 2023 2027 donc nous notre proposition, nous voyons que nous ne sommes pas les seuls, c'est simplement de supprimer cet article 16. Messieurs, vous C'est défendu, j'ajoute juste que les collectivités territoriales s'administrent librement, selon l'article 72 de la Constitution, il nous paraît donc utile et intéressant de supprimer cet article 16.

je suis dans une commune 64000 habitants, j'ai demandé à mon maire m'expliquer 2022, l'énergie, ça pesait 3 4 millions d'euros dans le budget 2023 c'est 7 millions d'euros.

Qui là se disent bah on est en train de regarder qu'on n'a pas une position commune parce qu'on ne va pas pouvoir faire le budget. Il y aura pas de capacité d'initiative voilà. Donc soit on asphyxie la capacité initiative des collectivités territoriales et et c'est le cas de cet article, excusez-moi mais moi je veux bien, ce qui a été dit tout à l'heure par Céline Bruel injuste. D'un côté on veut limiter à 0 5. On met sous tutelle, c'est ça que ça veut dire quoi donc je, je vous le dis, avec des mots pas plus fort que les autres que les autres, mais ça c'est attention parce que derrière, ça va se poser la question, certes, des services publics locaux des services rendus à la population. Mais on va avoir un problème de cohésion d'unité dans le pays, parce que si trop de collectivités territoriales et particulièrement les communes se retrouve en incapacité de se projeter dans les années à venir, mais dès 2023. a, on a un gros souci démocratique et un souci social hein. L'instabilité de désordres. Là l'avis de la commission sur ces trois amendements, monsieur le rapporteur général. C'est un avis défavorable en fait, je crois qu'il faut. Il faut essayer de, de tenir un cap. Je le redis, la majorité sénatoriale ne choisit pas forcément la facilité. Je dirais, en en en acceptant la demande ou la proposition du gouvernement de contenir ces dépenses mais d'abord, elle demande pour ne pas dire elle exige la réciprocité pour les dépenses de l'État et puis je crois et je pense aussi, je le disais tout à l'heure qu'un certain nombre de dispositifs notamment sur 2023 qui concerne le bouclier énergétique sur lequel nous aurons des exigences fortes parce qu'il s'agit sur des dépenses très qui qui pourrait être très élevé et que les collectivités locales ne pourrait pas supporter à elle seule, en totalité, c'est là où on doit avoir un niveau d'exigence, mais je dois dire que d'abord c'est un objectif, et deuxièmement, j'espère que ces difficultés ne dureront pas tout le quinquennat. En conséquence de quoi, de toute façon, il nous faudrait assez vite revenir et faire des choix ici et pour le redire : souvenez-vous de ce qu'est devenue la la programmation des finances publiques 2018, 2022 nous avions, nous avons demandé à plusieurs reprises des révisions et à chaque fois, le gouvernement nous a envoyé poliment sur les roses pour prendre une image qui en dit souvent plus long que de grands discours, donc un avis défavorable. Entendu, Monsieur le Ministre. Et merci monsieur le président. Autant je peux comprendre le débat, la controverse sur l'article 23 il viendra, même si je crois profondément que ça n'a rien à voir avec les contrats de Cahors, qui à l'époque, il avait été qualifié de mise sous tutelle, autant l'de Dell permet de prévoir de programmer de planifier les dépenses locales, enfin c'est pas quelque chose de nouveau qui est né avec cette loi de programmation des finances publiques, il existe depuis 2015. 2015, ça existe, donc voilà juste la question qui nous est posée, c'est ce qu'on veut être le seul pays d'Europe qui n'est pas capable de d'essayer de programmer de planifier, quelles seront les dépenses, l'évolution des dépenses dans les années à venir ou pas, tous les pays européens se dote d'un programme de stabilité dans lequel il prévoit, y compris les dépenses locales et leur évolution, il se dote d'une loi de programmation des finances publiques, c'est même une obligation pour bénéficier des fonds européens sur la relance et donc ils planifient programme voilà, en l'occurrence là on programme 31 milliards de dépenses supplémentaires. Pour les 5 années à venir pour les collectivités locales, ce qui est évidemment pas une Bremont ou une mise sous tutelle, on aura le débat sur l'article 23 et sur le mécanisme de sanctions que nous proposions dans le cas où la trajectoire serait pas respecté mais là en l'occurrence, on parle d'un ou de Dell, qui existe depuis 2015 et je ne crois pas qu'il y ait eu de mise sous tutelle des collectivités locales depuis qu'il existe un de Bon, donc nous avons 2 avis défavorable sur ces trois amendements que je mets aux voix monsieur Savoldelli souhaite et. Merci Monsieur le Président, juste sur le midi, j'en profite, à ma connaissance, la ville de Villejuif et toujours dans un contentieux sur le cadre du contrat de Cahors, malgré que ça soit la gauche qui est gagné aux dernières municipales et et l'engagement du contentieux est venue de l'ancien maire qui vous inquiétez pas, il avait pas beaucoup de changements, mais lui, qui était de droite, donc ce qu'est ce que vous me dites ce soir. Que l'état arrête tous les contentieux engagé vis-à-vis des collectivités qui étaient, qui sont encore dans des contentieux liés au contrat de Cahors, parce que si c'était pas bon, et si c'était pas juste. C'est pas la peine que l'État dépense de l'argent pour faire rentrer dans le rang des collectivités qui n'aurait soi-disant pas rentrer dans le cadre du contrat de Cahors, vous m'aurez dit oui, vous me dites non. Et on verra comment on fait après. Je n'ai pas d'autres explications de vote, donc je mets aux voix les trois amendements de suppression qui est pour. D'accord, qui est contre.

l'inflation la position qui vous est fait, monsieur le Ministre, c'est que l'objectif des d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est fixée au même niveau que l'inflation, donc voilà, ça permettra d'avoir des prévisions au plus juste.

L'avis de la commission sur ces deux propose d'accepter, on n'est pas tout à fait sur ce que j'appellerai cette indexation donc un avis défavorable. Le le gouvernement. Même avis pour les mêmes raisons. Très bien, donc je mets aux voix puisqu'ils sont différents, d'abord l'amendement Monsieur Féraud, qui est pour. Il n'est

Il n'est pas adopté ensuite un peu de concentration parce qu'il y en a six faisant l'objet d'une discussion commune nous commençons par un amendement 24 il y a la trois, qui sont identiques. qui est défendu par Monsieur la mairie qui a la parole. Oui merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues et avec votre autorisation, je peux présenter le 24 rectifié le 25 rectifié puisque c'est les mêmes même série d'amendements à l'initiative de notre collègue Arnaud Bazin et co-signé par beaucoup de nos collègues et il concerne les conseils départementaux et les préoccupations qui sont particulièrement importantes au niveau des conseils départementaux avec les problématiques sociales et qui concerne les Ayasse allocations individuelles de solidarité, ceux qui sont versés par les départements, notamment le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'apport et la PCH prestation de compensation du handicap qui seraient intégralement dans le Champ de ses dépenses réelles de fonctionnement. Et pour certains le représente, pour autant, environ 30 % du budget de fonctionnement des départements. Et l'amendement 25 rectifié donc dans le même esprit, à l'initiative de notre collègue Arnaud Bazin, il s'agit d'un amendement de repli et qui indique que, on l'état actuel du texte, les Hayes versée par les départements. Donc RSA a pas et puis Ch sera intégralement dans le Champ de ses dépenses réelles de fonctionnement, alors qu'elles ne peuvent pas de par définition être maîtrisé par les départements,

et 40 mais Marc Laménie a exposé les arguments comment mettre des contraintes sur des dépenses qui ne sont pas pilotable, et en particulier sur les allocations individuelles de solidarité donc le trente-neuf est un amendement de repli par rapport à la suppression de l'article, le quarante est un amendement de repli sur l'amendement de repli, je pense que il serait raisonnable de d'exonérer des dépenses absolument pas pilotable de contraintes qui s'exercent sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement des collectivités en particulier des départements. Madame Carrère maintenant oui merci 75 et peut-être aussi le second second volet. Oui non je rajouterai pas grand chose à ceux qui ont déjà dit, mes collègues juste un exemple : le contexte aujourd'hui et pas forcément favorable pour pour contraindre les collectivités locales dans leurs frais de fonctionnement, le département des Hautes-Pyrénées, au jour d'aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros en 2022 pour céder aux aux dépenses énergétiques et et les prise en compte des 3 points et demi d'augmentation du point d'indice et ça sera 20 millions d'euros en 2013 pour un petit département rural alors sortir les Hayes de ce cadre budgétaire parce que, comme l'ont dit mes collègues c'est ce sont des dépenses non-maîtrisées et non maîtrisable, je pense que cette une bonne, une bonne chose, je vous remercie et le deuxième hein manque demain est un amendement de repli, donc il a été défendu. Monsieur le rapporteur général sur ces 2 séquences. Alors je vais prendre les trois derniers 25 40 76 rectifié

ce qui facilite pour moi le la tâche puisque sur le 24 39 elles 75 rectifié, ce sera à chaque fois, une demande de retrait. Et le gouvernement. Oui. J'ai abordé tout à l'heure, la question de l'article 23 de la question de l'évolution des dépenses des collectivités locales et j'ai indiqué très clairement que les AIS. Ne sont pas des dépenses pilotables et qu'à ce titre-quand on parle d'un mécanisme de contraintes, il faut les retraités des dépenses dont on tient compte dans un mécanisme de contraintes et donc ces amendements me sens pour moi mal positionné, puisque c'est des amendements qui normalement devrait être présentés sur l'article 23 qui prévoyait, puisqu'il a été supprimé en commission, le cadre de contraintes pour les collectivités locales sur les dépenses de fonctionnement, prise en compte, c'était une demande très fort du président Sauvadet que dans le cadre de cet article 23 et du mécanisme de contraintes du pacte de confiance, il y a un retraitement des AIS j'des droits en disant que je serais favorable à des amendements qui retirent les AIS de ce pacte de confiance là en l'occurrence des amendements qui retraite les Hayes, de l'eau de Dell, mais le de d'elle n'est pas en lui-même une contrainte le Del c'est ce qui permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la progression des dépenses, donc c'est des un moment qui ont un sens, dans le cadre d'un mécanisme contraignant mais vous l'avez supprimé à l'article 23 et donc là, on se prive, vous êtes ben vous avez adopté un amendement de suppression en commission, je, je, vous, vous n'allez pas supprimer, vous allez peut être refusé de le réintroduire, parce que je vais le proposer avec un amendement du gouvernement mais en l'occurrence là ça n'a pas de sens, parce que le de Dell, il regarde l'ensemble de la progression des dépenses des collectivités locales

On peut pas dire que c'est totalement pilotable. Voilà et donc vous avez exclu les Hayes mais donc est-ce que ça veut dire que vous considérez que les fonds européens, des régions, ces pilotes pilotable voyez, c'est pour ça que sur le mécanisme pacte de confiance mécanisme contraignant ma proposition au départ, c'était que on retraite, on choisit les dépenses qu'on retraite et qu'on le fasse par décret après concertation avec les collectivités locales, mais s'il y avait des amendements sur les Hayes, j'étais prêt à être favorable mais là en l'occurrence, ça veut dire que tout le reste sont des dépenses pilotable or, c'est pas le cas, donc moi je pense qu'il faut garder le de Dell telle qu'il existe aujourd'hui et depuis 2015, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses des collectivités locales, s'il y a mécanisme de contraintes à ce moment-là, retraité des dépenses les Hayes parce qu'elle a d'autres qui peuvent être retraités mais là, avec ces amendements de facto le message que vous envoyez, c'est que toutes les autres dépenses des collectivités locales, sont pilotable puisqu'elles ne sont pas retraités comme les AIS, moi je considère pas ça, donc avis défavorable. Madame vous vouliez ajouter un mot. Monsieur le Ministre, on ne peut pas être d'accord avec vous. L'article parle d'un objectif de réduction des dépenses publiques, les monte un sens un objectif de réduction des dépenses publiques, c'est de ça dont il est question et on ne peut pas demander à un département qui verrait par exemple le nombre de ses bénéficiaires du RSA pour des raisons complètement indépendante de sa volonté, être pénalisés au regard de cette et cet objectif c'est cela dont on parle, et donc on ne peut pas être d'accord avec ce que vous venez de dire. je je commence par consulter le Sénat sur les nous amendement 24 39 et 75 sont identiques et qui ont fait l'objet d'la vie d'une demande de retrait du rapporteur général, quels sont ceux qui sont pour.

je compte les contres là. ensuite des amendements donc 25 E 40 et 76 qui ont fait l'objet d'un avis de sagesse ou favorable du rapporteur général et d'un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Contre. Ils sont adoptés, l'article 16. Qui est pour,

Merci Monsieur le Président, c'est un amendement qui reprend une proposition du rapporteur général de l'Assemblée nationale et qui visait engager les collectivités locales à adopter un budget Vert d'ici la fin du quinquennat il vise à déployer le budget vers des collectivités, l'année suivante de l'adoption de la nouvelle nomenclature de comptabilité publique, M. 57 qui sera adopté le 1er janvier 2024 il rehausse également le seuil de dépenses total de 50 à 100 millions d'euros, cette mesure contribuera à accélérer la transition écologique en intégrant au modèle économique la qualification des dépenses, eu égard à leur impact climatique. C'est une une demande de retrait, moi je pense que la la démarche être aujourd'hui à ce stade prématuré, j'observe d'ailleurs qu'il a eu, il y a pas eu de concertation avec les élus pour tenter de se mettre d'accord, je note également que la méthodologie qui est appliqué aux dépenses de l'État, elle n'est pas forcément duplicable en l'état aux collectivités et il me il me paraît qu'il faut travailler sur la méthodologie de du fameux. Budget environnementale avec les collectivités, je veux rappeler que dans le PLF pour 2023 sur les 570 milliards d'euros de dépenses budgétaires et fiscales 416 excusez du peu, sont considérés comme neutres. 94 ne sont pas cotées et donc il en reste 59 milliards côté favorable, défavorable ou mixtes, c'est-à-dire à peine plus de 10 pour 100 des dépenses totales les départements concernerait toutes les régions et départements mais seulement 115 communes et 107 EPCI, j'ai regardé de près l'objet de l'amendement, mais cette aussi plus de 40 % des dépenses totales du bloc communal, la question que je pose et que je ne nous pose aujourd'hui et ce qui nous paraît nécessaire d'ajouter à ce stade des contraintes administratives et comptables relativement lourde pour arriver à ce type de résultats, d'où la demande de retrait. Oui, quand on a rencontré les associations d'élus avec Christophe Béchu et Caroline Cayeux, toutes les associations d'élus nous ont fait part de leur intérêt à faire en sorte, hein, que les collectivités locales les plus importantes puissent adopter un budget vert et de à ce qu'on travaille avec les associations d'élus à ce qu'on ait un référentiel commun, État, collectivités locales, c'est objectivement utile pour savoir exactement où va la dépense publique dans notre pays, quelle que soit la dépense publique, qu'elle soit de l'État ou de des collectivités locales pour savoir ce qui est favorable à l'environnement, ce qui est défavorable à l'environnement, donc c'est un amendement effectivement d'initiative parlementaire, qui prévoit un budget Vert pour les plus grandes collectivités au-dessus de 100 millions d'euros, je pense que l'essentiel parce que la réalité c'est que je pense qu'aujourd'hui la plupart de ces collectivités, en tout cas un grand nombre d'entre elles se sont dotés d'un budget Vert mais derrière budget Vert il y a beaucoup de collectivités qui mettent des choses très différentes et pas la même cotation pour les mêmes dépenses par la même prise en compte des dépenses, ce qui serait utile pour qu'on ait une vision exhaustive à l'échelle nationale, c'est qu'on ait un référentiel commun qu'on va construire avec les associations d'élus, donc moi je suis favorable à cet amendement juste répondre au rapporteur général parce que on fait souvent la critique sur dans le budget de l'État, il y a plein de dépenses qui sont non coté on sait pas si favorables ou défavorables, bah oui, j'ai envie, dire et puis heureusement il y a notamment le salaire des fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires les allocations sociales, heureusement qu'on ne va pas regarder ce que font les gens de leur salaire ou de leur retraite ou de leurs allocations sociales si elles font des dépenses avec leur argent, qu'elles ont gagné favorables ou défavorables à l'environnement, là pour le coup on basculerait dans un autre type de régime auquel je suis pas totalement favorable et donc oui, il y a de toute façon une part des dépenses publiques qui ne pourront jamais être côté parce que c'est ce qui permet de faire verser un salaire aux fonctionnaires une retraite ou des allocations sociales.

et qu'aujourd'hui un cadre a été édictée par l'Association des maires de France France urbaine et forcit qui en fait prend la maquette, M. 57 prend des dépenses et les projets et ça donne un résultat qui est là, je rejoins le début du propos du ministre est complètement inexploitables parce qu'en fait une grosse partie des dépenses dépenses de ces collectivités ne sont pas classifiées typiquement toutes les dépenses de personnel en gros 50 % de la dépense quand on regarde les sections la section d'investissement, on a en gros 20 % des dépenses d'investissement qui sont cotées, elles sont toutes cotées comme étant réputée favorable à l'un à l'environnement puisque dès qu'on fait des travaux dans les bâtiments publics le présupposé est que la dépense est favorable à ce qu'on vient améliorer le bâtiment donc on vient améliorer ses performances thermiques et je vais vous le dire, ici les dépenses qui sont considérés comme défavorables, ce sont les dépenses informatiques aujourd'hui, peut-on dire que toutes les dépenses informatiques sont défavorables à l'environnement donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui ce cadre effectivement il existe, il est complètement perfectible, donc quel va être le sens de venir demander aux collectivités de faire quelque chose qui est simple à faire, qui va pas mobilisé beaucoup de temps, mais moi je pense qu'il y a un document qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant, c'est le rapport sur le développement durable, qui est présenté juste avant le débat d'orientation budgétaire de ces collectivités qui permet, au-delà des chiffres, de présenter des politiques publiques et la politique en matière de développement durable est par nature une politique transversale et au-delà des seuls enjeux qui se matérialise par des euros, c'est parfois des choses qui sont dans des actions que fait la collectivité et pour lesquels il est assez difficile de dire si ces 5, 10, 15 ou 20 euros ou qui a affecté donc pour ces raisons-là, moi je suis plutôt défavorable à cet amendement, puisqu'en fait, dans les faits, il existe déjà mais il est complètement inopérant. Monsieur voyez. C'est une explication de vote on on s'abstiendra, parce que nous nous pensons nécessaire et la plupart des collectivités s'engagent à évaluer leurs leurs à s'interroger, comme vient de le dire, ma collègue avare d'ailleurs sur les outils de la transversalité qui permettent de de s'engager dans cette transition, il n'empêche que je crois que nous devons défendre ce principe d'être capable d'évaluer pour les collectivités avec elle et avec une élaboration avec les collectivités elles-mêmes ce que sera demain des des Budgets vers de collectivités, donc nous ne voterons pas cet amendement parce que nous pensons que la concertation est aujourd'hui nécessaire, on appuie sur les premières expériences menées par ces collectivités les Tu le rapporteur général. Oui, je vais ajouter quelques mots qui finalement s'inscriront à la fois dans l'intervention du sénateur briller et de Christine Lavarde je pense que Christine Lavarde a parfaitement raison le ce document cette présentation du rapport de développement durable est obligatoire depuis, je pense à peu près une décennie, il a fallu un certain temps, puisque là non plus, il y a pas forcément de méthodologie, moi ce qui me préoccupe le plus, monsieur le Ministre, le gouvernement 7 enorgueillit de nous présenter depuis 2 ans déjà, à budget Vert, j'ai toujours émis un certain scepticisme et je crois que le gouvernement m'a donné raison, nous a donné raison, en tous les cas sur les sceptiques, puisqu'à peine le 1er, gouvernement de la nouvelle Première ministre, installé, vous avez le gouvernement a fait appel à à une mise en condition pour changer, finalement, de rythme et de logiciels en invitant la Nancéienne Valérie Masson-Delmotte et ses équipes à venir faire oeuvre utile de pédagogie et j'espère plus pour inculquer les enjeux, les préoccupations environnementales, écologiques, alors c'était bien la peine de nous faire je dirais beaucoup de volume sur ce sujet-là et je prendrai, je l'ai dit tout à l'heure un 2ème exemple qui n'est pas dans la sphère publique, qui est dans la serre privé ce que j'ai tout à l'heure quand je vois aujourd'hui que la BCE finalement met un carton jaune aux banques en leur disant : sur la finance verte, il y a une nécessité à ce que le secteur bancaire prenne à bras corps et véritablement ses préoccupations pour que soit porté et accompagné la nécessité un peu de changer le logiciel de développement de nos économies pour les Verts, dire vraiment, voilà, je pense que, au-delà de l'affichage, il faut des actes et puis et enfin je pense que pour ces réflexions, il faut aussi amener un peu de diversité d'opérateur pour trouver les bonnes méthodes, je crois et je respecte beaucoup, l'institut pour le climat, mais je pense là aussi que, un peu de compétition interne sur des compétences avérées ne nuirait pas à la progression de la prise en compte de ces sujets Donc nous allons nous prononcer sur cet amendement 57 qui, il y a donc un avis favorable hein du de la commission 57 c'était un avis favorable.

Alors attendez qu'est ce que j'ai dit une erreur le le la l'avis de la commission était favorable, défavorable et et j'étais en train de compter les pour. Et le gouvernement est favorable, donc il est pour cet amendement. D'accord, qui est contre, il y en a un peu plus et donc il n'est pas adopté à l'article 17 nous avons 2 amendements de suppression identiques et nous commençons par le groupe socialiste, Merci monsieur le président, donc le présent amendement vise à s'opposer à ce qui s'apparente à une nouvelle contraction des moyens réels de la sphère sociale sans tenir compte des leçons de la pandémie du Covid 19 dans la loi de programmation, dit le PLFSS 2023 cette contraction se traduira par un déficit ramené à 6,8 milliards contre 24,3 milliards en 2021 et de or de 17,8 milliards en 2000 et un Ondam hors dépenses qui a la crise sanitaire, en hausse de 3 7 % contre 5,4 pour 100 en 2022 soit largement inférieur à l'inflation. Et ce alors même que nous connaissons une crise hospitalière aiguë en matière notamment d'accès aux urgences, il est dès lors proposé de s'opposer à cette orientation qui ne tirent en rien les des leçons des erreurs du passé. le groupe CRCE Monsieur Mathieu. Merci monsieur le président, comme vient de le dire, mon collègue, l'article 7 prévoit une hausse des dépenses de santé inférieur à l'évolution naturelle des dépenses estimées par la commission des comptes de la Sécurité sociale de plus 4 % une hausse des dépenses du budget de santé inférieur au taux d'inflation, le gouvernement prévoit ainsi que les dépenses des hôpitaux progresseront de 4 virgule 1 % en 2023, de 9 % en 2024 et de 8 % en 2027 autrement dit : non seulement le gouvernement ne prévoit pas d'augmenter le budget des hôpitaux dans l'ensemble des indicateurs sont déjà dans le rouge, comme par exemple le dernier en date, les urgences des urgences pédiatriques mais Pierre, il prévoit de réaliser des économies sur le dos de la santé de ces prochaines années, cette logique austéritaire qui a démantelé le service public hospitalier ces 30 dernières années seraient donc poursuivies et amplifiées avec ce cadre pluriannuel, ce que nous refusons pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de certains articles dont les conséquences seraient irrémédiablement de nouvelles fermetures de lits d'hospitalisation et d'hôpitaux de proximité sur leur territoire. L'avis de la commission sur ces deux amendements monsieur rapporteur général. C'est un avis défavorable, notre collègue sénateur, je pense que le propos est un peu excessif, mais je vous laisse, je vous en laisse évidemment la liberté, je veux simplement quand même rappeler que ces objectifs font partie de la vie politique obligatoire dans la loi de programmation, en application d'ailleurs de la loi organique et que le rôle de cet article, finalement, c'est de pouvoir permettre au Parlement de vérifier chaque année lors de l'examen du PLFSS à quel endroit se trouve par rapport à cette trajectoire et donc d'une certaine manière, c'est un suivi et c'est aussi une évaluation. Avis du gouvernement. Défavorable. Merci. Je mets aux voix c'est d'amendement de suppression qui est pour. Qui est contre et ils ne sont pas adopter vient ensuite un amendement 70 du gouvernement que le ministre présente. Oui, c'est un un amendement de retour au texte initial, qui prévoyait une programmation dont dame jusqu'à 2025 donc sur 3 ans, là où la commission des finances, a ajouté 2 années, 26 et 27 par cohérence avec ce que vous avez voté tout à l'heure à l'article 12 sur les crédits du budget de l'État sur 3 ans, il nous semble préférable de rester sur 3 ans également pour le Honda. La ville de la commission sur l'amendement 70, monsieur le rapporteur général. inscrive comme d'abord la commission Affaires Sociales a proposé 2000 26 et quand on arrive à faire 2026 moi je j'invite le gouvernement à faire également sur la période de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2027 un avis défavorable. Entendu. L'amendement le je mets aux voix l'amendement 70 qui est pour.

nous demandons la suppression de cet article, puisque celui-ci encore des dépenses de la gestion administrative des régimes obligatoires de les bases de la sécurité sociale mais aussi l'établissement d'euros de retraite additionnelle de la fonction publique, on a eu ce débat il y a peut-être à peu près une heure ou une heure et demie sur les emplois, les conventions d'objectifs et de gestion de la sécurité sociale, le bilan déjà est dramatique, 2018 à 2022 900 emplois ont été supprimés dans les ça 8000 dans les CPAM. 1150 dans les Urssaf et entre 2000 et 3000 estimés dans les caisses d'allocations familiales. Donc à tout cela s'ajoutent les 20000 emplois qui ont été supprimés entre 2009 et 2017, donc là, pourquoi nous demandons la suppression de l'article parce que nous contestons le bien-fondé de la trajectoire qui est proposé, qui va encore se traduire par une trajectoire de encadrement qui va faire une diminution, ajouté au vote que une partie d'entre nous ici on eu pas cette partie-là, mais vous avez tout à l'heure, voter la suppression de 125000 emplois, hein, et bien d'accord. Avis de la commission sur cet amendement de suppression. Alors un avis défavorable je vais je vais redonner quelques éléments d'explication à notre collègue le sénateur Savoldelli alors la présente loi de programmation fixé un objectif de diminution des dépenses de gestion administrative des caisses de Sécurité sociale. De un virgule ces dépenses en fait ont baissé de, de 2 % par an de 2018 à 2020 et ensuite en raison de la crise sanitaire, le mouvement a été stoppé le gouvernement à proposer un objectif là de stabilisation pour les 5 années qui viennent, compte tenu de l'inflation. Je vous informe et vous le savez que sur la proposition de la commission affaires sociales nous avons précisé qu'il s'agit bien de ne pas dépasser le ratio actuel, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, la poursuite des efforts possibles. D'optimisation des dépenses de gestion et donc il n'est pas souhaitable d'abandonner un objectif de maîtrise des dépenses administratives comme le proposent les auteurs de l'amendement en supprimant l'article.

Qui est contre, il n'est pas adopté, hé bien, ensuite, un amendement du gouvernement, le numéro 71 Monsieur le Ministre. C'est un amendement quasi rédactionnelle qui va dans le sens de ce qui est souhaité, je crois, par les sénateurs, et notamment la sénatrice Doineau

Si c'est un si c'est un avis de sagesse, Monsieur le Ministre. Entendu donc sur l'amendement 71 du gouvernement avec sagesse de la commission, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, il était adopté et nous passons à l'article 18 dans le sang, ensemble, qui est pour.

Merci monsieur le Président notre amendement c'est un amendement de suppression de l'article 19 cet article 19, il prévoit une mise en réserve en début d'exercice d'au moins 0,3 pour donc de 2 choses l'une : soit cette disposition, elle a pour but de pouvoir annuler des crédits budgétaires dans le cadre de l'Ondam décider, soit elle a pour but de pouvoir faire face aux crises en fin d'année, notamment de l'hôpital comme on connaît en ce moment sur la pédiatrie crise due à l'insuffisance de l'Ondam lui-même prévu par l'article, mais dans les 2 cas, il y a quelque chose qui cloche et d'ailleurs, une telle disposition n'existait pas dans la loi de programmation des finances publiques précédentes, donc notre proposition est très simple, c'est de supprimer l'article 19. Messieurs Savoldelli même. Oui, merci Monsieur le Président, Clovis, mes chers collègues. Je mets à votre crédit que ces mises en réserve prudentielles de crédit, elles ont été mises en place en 2010, donc on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de l'exécutif actuel. il y a des précédents. Et il y a tellement de précédents que ça a été étendue en 2015, aux activités de soins de suite et de réadaptation et psychiatrie. Val-de-Marne 2ème, département de la PHP et cetera, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais ça représente un montant de 412 millions d'euros en 2017 415 millions d'euros en 2018 et en 2019 chaque année 0 3 % des crédits pour la santé sont mis en réserve et débloqué en fin d'année, et là c'est pas seulement la vie de notre groupe. Pourquoi on demande la suppression de cet article, parce qu'on a bien lu les résultats de la commission d'enquête du Sénat sur la situation de l'hôpital. Et la commission d'enquête du Sénat la dénoncer, système de mise en réserve d'une partie du budget des des hôpitaux. Donc, on essaie d'être cohérent entre notre travail collégial qui des fois peut même faire unanimité et le de traduire par un amendement et là l'amendement c'est la poursuite du travail sénatorial qui a mis en exergue que la mise en réserve des Budgets des hôpitaux mise en énerve était complètement irresponsable, là de ce coup-ci. L'avis de la commission sur ces deux amendements de suppression, monsieur le rapporteur général. C'est un avis défavorable, effectivement, le sénateur Savoldelli a bien fait de rappeler que c'est un dispositif qui existait depuis 2010 mais ça c'est le travail collégial de de ceci étant la mise en réserve ne signifie pas l'annulation puisque ça permet aussi de gérer les risques de dépassement. Sur la base, en particulier les avis du comité d'alerte du respect de l'Ondam auquel la loi a confié cette fonction, je souligne que, sur proposition de la commission des affaires sociales, il a en outre été précisé que la mise en réserve doit concerner toutes les composantes de l'Ondam et, à ce stade, il ne me paraît donc pas souhaitable de se priver de cet outil qui doit contribuer parmi d'autres d'ailleurs, à participer à mieux maîtriser l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Très bien. Qui est pour ces 2 amendements de suppression. Quels sont ceux qui sont contre. Ils ne sont pas de noter et nous avons ensuite l'amendement 72 du gouvernement que le ministre présente. Oui, comme les amendements précédents c'est un amendement de rétablissement du texte initial à nouveau pour prévoir l'Ondam sur 3 ans au lieu de La avis du de la commission, monsieur le rapporteur général. Lors. Quels sont ceux qui sont favorables à cet amendement, quels sont ceux qui sont pour cet amendement du gouvernement avec avis défavorable de la commission. Pour. Pour. Abstention est pas adopté et donc nous nous prononçons sur l'article 19 qui est pour.

merci Monsieur le Président, aux exonérations de cotisations sociales même même antérieure à la la présente loi, il demande ainsi au gouvernement de proposer pour chaque dépenses sociales existantes, une date d'extinction avant 2030, les délais qui sont laissés au gouvernement, plus d'un an et demi d'analyse pour une mise en application progressive jusqu'en 2030 permettront de ne pas modifier d'une manière trop brutale, le cadre existant. Qu'avait de la commission sur en général. C'est une demande de retrait depuis la loi organique de du 14 mars 2022, l'évaluation des niches sociales et prévue annuellement pour au moins un tiers d'entre elles dans le cadre du projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale de l'exercice clos la première évaluation doit donc intervenir d'ici à juin 2023 et chaque mesure devra faire l'objet d'une évaluation, une fois tous les 3 ans, j'ai donc le sentiment que ça satisfait largement le 1er objectif de l'amendement, l'amendement 14 prévoit en outre la suppression de toutes les mesures d'exonération avant 2030, cela me semble-t-il, préjuge des conclusions de l'évaluation que d'ailleurs vous demandez les dispositions de la loi organique me paraissent à ce stade, plus pertinente. L'avis du gouvernement. Oui défavorable propose d'en rester à l'équilibre retrouvé dans la dernière révision de la loi d'organiser la loi organique sur les lois de financement de la Sécurité sociale. Je mets aux voix donc cet amendement numéro 14 avec double avis défavorable qui est pour. Qui est contre, abstention, il n'est pas adopté, nous votons sur l'article 20 qui est pour l'article 20. Qui est contre, il est adopté à l'article 21 nous avons à l'amendement numéro 49 de monsieur Savoldelli. Qui est défendu sur lequel la Commission a une opinion et et le gouvernement là même donc. Je me vois cet amendement 49 avec double avis défavorable qui est pour. Il est contre, n'est pas adopté, nous avons l'amendement 74 du gouvernement que le ministre présente. Oui, très rapidement, vous avez précisé en commission des finances, le cadre de l'évaluation de la qualité de la dépense publique, vous avez ajouté 3 éléments hein, liste la liste des évaluations transmises au Parlement, s'est satisfait puisqu'il y a une disposition qui a été adoptée dans le PLF adoptée aujourd'hui enfin réputé adopté sauf motion de censure contraire dans le 49 3 un amendement qui a été retenue et donc cette liste d'évaluation est satisfaite par la disposition que qui a été introduite en PLF de la publication de l'ensemble des données, ça pose des sujets de droit de secret fiscal de secret des affaires évidemment transmettra toutes les données utiles dès lors que c'est juridiquement possible et trois la liste de l'ensemble des personnes auditionnées un droit de réponse pour les personnes ou les organismes concernés ça pour le coup, on propose de le garder, qui est un ajout de la commission, pour la liste des évaluations s'est satisfait par le PLF pour la publication des données, ça pose un vrai problème de droit et de secrets notamment secret fiscal et secret des affaires, donc on propose de revenir juste sur ces 2 dispositions dont une est satisfaite.

ceci étant, je ne vois pas bien l'intérêt que le principe de publication de la liste des dites évaluation soit prévue par la loi de finance, mais bon, sur le second point, vous mettez en avant des incertitudes juridiques qui entourent la publication des données, il me paraît que dans la mesure où les données couvertes par le secret sont exclus explicitement du Champ de la disposition, je vois mal à quelle incertitude juridique, le gouvernement pourrait faire face, enfin, j'observe que le gouvernement n'a pas respecté les récentes évolutions de la LOLF, qui prévoit que les documents budgétaires doivent être mis à disposition du public dans un format largement réutilisables, en d'autres mots, sous forme de tableur voilà une disposition adoptée par la commission des finances vous y invite donc à nouveau un avis défavorable, comme je l'ai dit dans mon propos introductif en forme de commentaire. Je mets aux voix cet amendement du gouvernement avec avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il est pas adopté, je soumets l'article 21 au Sénat qui est pour l'article 21 qui est contre, il est adopté, je mets aux voix, l'article 22 mai votre. L'article 23. Il fait l'objet d'un amendement qui a été supprimé, elle fait l'objet d'un amendement du gouvernement, l'amendement 73, monsieur le Ministre. en réalité, on en a beaucoup débattu beaucoup parlé depuis le début de l'examen de ce texte dans la discussion générale, à l'occasion de différents amendements, donc je vais être bref, c'est un amendement qui est pour nous le pendant de l'eau de Dell, que vous avez voté tout à l'heure, si on veut fixer un cadre crédible d'évolution de la dépense publique pour les collectivités locales, il faut prévoir un mécanisme d'encadrement, j'ai dit dès mon intervention liminaire. Que je pense que le plus probable est que ce dispositif n'est pas à être actionnés utilisé parce que les collectivités locales sont parfaitement consciente aussi de leur rôle dans la maîtrise des dépenses publiques et d'ailleurs, elle nous l'ont dit, quand on a échangé avec les les associations d'élus, pour certaines, elles l'ont écrit notamment l'association des départements de France, qui ont dit qu'il. Pouvait tout à fait concevoir de tenir la trajectoire fixée modulo que les AIS en soit sorti, c'est pour ça que j'ai donné un avis favorable dans l'article 23 pour les sortir les les intercommunalités de France on dit que ce dispositif : pas de pacte de confiance sortait complètement la logique Cahors il y avait il y a des raisons de rétablir cet article 23 parce qu'il permet de fixer un cadre voilà et donc de donner aussi de la crédibilité à la trajectoire que nous adoptons pour autant je suis lucide sur le peu de chances que cet amendement soit adopté au regard des différents votes qui ont eu lieu ce soir mais il me semble important de vous le reproposer et qui sait, peut-être à la toute fin de ce texte peut être que nous aurons un à un vote favorable, en tout cas je le souhaite. C'est. Principe des trompettes de Jéricho, monsieur le rapporteur général. Oui, j'ai entendu quelques sourires et même un peu plus Monsieur le Ministre dans votre à la fin de votre propos, Vous savez, je ça échaudé craint l'eau froide quand même rejetée à l'Assemblée nationale, rejeté au Sénat, c'est plutôt mal vous persistez, vous signez, c'est parfaitement votre droit je voudrais peut-être en quelques mots vous dire d'abord ce qu'on rejette, c'est finalement la méthode d'un gouvernement qui s'est engagé à tourner la page des contrats dits de Cahors pour finalement les rétablir et je dirais même les rétablir empire il y a des pans entiers de l'Arctique, qui sont un vilain copier/coller. Des contrats de Cahors, qui figurait d'ailleurs dans la presse dans notre programmation et je vous invite à le vérifier, c'est juste un peu consternant alors la principale innovation, elle consiste à ras, une approche des catégories de collectivités, vous savez, les fameuses strates, moi je dis c'est stratosphériques. En tous les cas je j'ai le sentiment que de vouloir prendre des bouts des catégories pour expliquer comment une strate permettrait ou des collectivités d'une strate mais pas d'une autre, enfin souvent ça reste bien complexe, enfin l'exclusion des dotations pour les collectivités qui dépasserait l'objectif me paraît complètement inacceptable puisque, quand même, à partir de quand on attente à la libre administration des collectivités territoriales, je pense qu'on peut travailler en bonne Intelligence, vous évoquez en permanence les discussions avec certaines associations qui ne nie pas qu'il y a des efforts à faire, je crois que depuis le début de cette séance publique nous portons également dans un même esprit de responsabilité, la participation à un effort, mais je ne vois pas que le dispositif que vous proposez avec cet article 23 soit un changement de méthode, à défaut, dit radical qui nous permettent de regarder avec davantage d'optimisme l'avenir et vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, Cahors, on a vu ce que ça a donné beaucoup appellent le dispositif que vous proposez là Cahors bis et pour l'instant, vous l'avez compris ici au Sénat, nous n'en voulons pas.

je pense, je ne vais pas tort, il y a une volonté de mise sous tutelle des collectivités territoriales à tard à travers votre volonté de réintroduire l'article 23 que unanimement ici, nous demandons la suppression. Monsieur Bruillet souhaite aussi, c'est expliquer son vote pour n'explique. Question de vote pour dire bien sûr que le besoin d'encadrer les collectivités n'est pas sain, il faut aussi, il y a des réformes de structure à faire augmenter la décentralisation faire confiance les laisser, elles ont la règle d'or, elle ne génère pas de déficit, je pense que notre pays sera bien inspiré d'être un peu moins jacobin et un peu plus attentif à l'autonomie des collectivités territoriales. Donc je mets aux voix cet amendement du gouvernement avec avis défavorable de la commission qui est pour. Hé bien, qui est contre. Il n'est pas adopté et donc on en reste à l'amendement 23 supprimer. Je vais mettre aux voix l'amendement 24. Qui est pour.

Je dois maintenant mettre aux voix l'ensemble du projet il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Une fois deux fois Monsieur Bruillet. quelques explications, malgré l'heure tardive, chers collègues, nous avons dans cette séance supprimé par un amendement de la majorité sénatoriale 125000 emplois il y a de nombreux services publics qui sont en grande souffrance, nous n'avons pas dit quelles seraient ces emplois supprimés malgré la demande d'ailleurs du ministre de précisions sur ce sujet, mais je dois dire que cet amendement suffirait à lui-même à annihiler les progrès qui ont pu être obtenus, je pense notamment à la suppression de l'article 23 ou à quelques amendements de second rang au plan écologique, plus simplement, le Sénat s'il a supprimé l'article 23 qui était sans doute un contrat mais pas du tout un contrat de 2 confiance à tout de même maintenu l'article 16 qui est une trajectoire de contraintes des collectivités, ces considérations, chère collègue qui, évidemment, nous voterons contre ce projet de loi de programmation qui au fond à vue des fiançailles, parfois un peu houleuses entre le projet gouvernemental et le projet de la majorité sénatoriale, je ne suis pas sûr que l'Union ainsi soit bénéfique à l'ensemble des des collectivités et des citoyens de notre pays. où l'examen de ce texte, ça a démarré ce soir, nous nous étions devant un choix décisif devant engager notre responsabilité pour les les 5 années qui viennent et, en cela c'est c'est même de l'avenir de notre pays et de ses de ses finances que nous devions discuter la majorité sénatoriale voulait nous faire la démonstration ce soir que l'effort n'était pas suffisant, mais hélas, nous avons pu constater, elle a fait la démonstration qu'elle quand elle est plus loin, mais pour une trajectoire plus ambitieuse, mais elle nous a pas démontré comment elle pouvait on pouvait aller plus loin en matière de de réduction des dépenses publiques, par ailleurs, je pense que le le rejet de nombreux amendements de de rétablissement du gouvernement ben tout nous incite à à nous abstenir sur ce texte, merci. Monsieur sont tard a demandé d'expliquer son vote. Oui, merci Monsieur le monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, dans quelques minutes, le Sénat se prononcera sur la trajectoire budgétaire de notre pays pour les 5 ans né à venir, il s'agit de la 6ème loi de programmation des finances publiques depuis la révision de l'Arctique 34 de la Constitution, nous avons donc désormais un peu de recul sur cet exercice, l'expérience nous montre que, malheureusement, aucune loi de programmation n'est respecté, au-delà du fait des crises que les crises surviennent régulièrement, nous constatons que, même dans les périodes épargné par ces crises, je pense par exemple aux années 2012 à 2018 la trajectoire n'est pas respectée, il risque hélas d'en être de même pour la période 2023 2027 au-delà même des forts aléas conjoncturels pesant sur les années à venir, nous avons dénoncé une trajectoire beaucoup trop optimiste et donc irréaliste, c'est la raison pour laquelle le Sénat a voté une trajectoire de redressement des comptes plus ambitieuse en proposant que l'État fasse davantage d'efforts d'économies à hauteur de ce qu'il demande aux collectivités territoriales, cette trajectoire telle que nous l'avons modifié permettra un retour sous les 3 % de déficit dès 2025 plutôt que de 1027, rappelant que tous les autres pays européens ont prévu d'y revenir ou d'y parvenir en 2025 au plus tard, l'Italie et l'Espagne et la Grèce même dès 2023 en moyenne le déficit public en Europe serait de moins de 2 % en 2025 et de 1 pour 100 en Allemagne, par ailleurs, si les collectivités doivent participer à l'effort de redressement des comptes, nous nous sommes opposés au pacte dit de confiance proposé par le gouvernement, car il s'apparente en réalité à un acte de défiance envers les élus locaux qui prévoyait, contrôles et sanctions contraires à la libre administration des collectivités territoriales, rappelons qu'une règle d'or s'applique déjà au budget de fonctionnement des collectivités locales et qu'elles dégagent un excédent budgétaire et ne pèse donc pas sur le déficit public et très peu sur la dette ainsi modifié par notre Haute assemblée le projet de loi de programmation des finances publiques dans notre pays a besoin recevra l'approbation du groupe, les républicains, je vous remercie. merci Monsieur le Président groupe socialiste comme je crois l'ensemble des groupes du Sénat, se réjouit de la suppression de l'article 23 et du fait que notre assemblée écarte ce dispositif dont nous considérons qu'il s'apparente à une mise sous tutelle des collectivités territoriales, pour autant, nous ne voterons évidemment pas ce cette loi de finance cette loi de programmation des finances publiques parce que nous ne nous retrouvons pas du tout dans le cadre qui est défini ni par le gouvernement, ni par les modifications qui ne sont pas si considérable que cela d'ailleurs de la majorité sénatoriale, j'ai d'ailleurs entendu l'explication de vote de notre collègue Didier Rambaud il ne conteste pas la trajectoire que nous ah que nous que vous allez voter ce soir sur les finances publiques parce qu'elle ne serait pas souhaitable, mais simplement parce qu'elle ne serait pas possible pour nous, nous considérons par ailleurs qu'elle n'est pas souhaitable pas souhaitable et que cette loi de programmation, même si je sais qu'elles ne sont jamais respectés, elles ont quand même de l'importance, elle ne permet pas de dégager les ressources dont notre pays aura besoin pendant le quinquennat alors nous savons l'importance d'une loi de programmation des finances publiques, tout le monde a vu qu'elle n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, d'une certaine manière, tout commence ce soir pour cette loi de programmation des finances publiques, nous, pour notre part, nous ne nous reconnaissons pas dès le départ dans le projet, qui maintenant va faire l'objet d'une discussion, je n'imagine très nourris et très riche, entre le gouvernement et les républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avais évoquée au tout début, dans la question préalable : la question de la des programmation des finances publiques. On y On y est on a abordé trois enjeux importants hein, toutes les administrations centrales publics, les collectivités territoriales et de la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on y passe des heures, mais c'est pas des heures perdues, hein, c'est des questions essentielles, et on a pu assister par rapport au projet initial à une surenchère de la majorité sénatoriale. ça a été évoqué 125000 emplois. Public. On peut discuter à la marge. Mais la plupart de ses employes à chaque emploi c'est un service public, donc il va falloir supprimer des services publics. vient de c'est c'est ça qu'on nous propose de voter. Autre omission quand même dans les conclusions de cette affaire. C'est que la si ont voté pour la loi de programmation avec les surenchères de la majorité sénatoriale. on va voter ce qui vont voter pour vont voter une perte de 2009 milliards pour les collectivités territoriales. ça va être dur à expliquer ça, quand on revient dans son département dans ces villes. De dire qu'on a été dans une alternative qu'on a essayé de faire progresser la loi de programmation initiale en disant: oui d'accord mais on a quand même voté, moins de 9 milliards pour les collectivités territoriales, on est très soucieux de la libre administration des collectivités territoriales, donc voilà, tout cela va être caduque, je vous avoue que je me suis demandé dans les heures passées et dans les allers-retours avec ses votes importants hein 125000 emplois, moins de 9 milliards pour les collectivités territoriales, je me suis dit : mais, attends, Pascal, est ce que tu es pas en train d'assister à un nouveau pacte de gouvernement. Je me suis posé la question. On aura sûrement la réponse dans les semaines à venir, en tout cas le groupe communiste votera contre cette loi des des bras mation des finances publiques. Je n'ai plus de demandes d'explications de vote une fois deux fois donc je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 qui est pour. Qui est contre. Il est noter. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance, jeudi 3 novembre à 10 heures 30 pour l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables, la séance est levée.

Merci